est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

Pourquoi, madame la ministre, nous avoir présenté ce texte ? Après une semaine de débat ici, nous ne comprenons toujours pas votre objectif. Vous affichez, dans vos discours et vos écrits, votre volonté de maîtriser l'immigration, d'améliorer le droit d'asile et de réussir l'intégration. Très bien Nous vous avons écoutée pendant une semaine, vous-même ou M. Collomb, et nous ne comprenons toujours pas ce qui correspond à vos objectifs dans votre projet de loi. Ce texte est même contre-productif à plusieurs titres : d'abord, à cause de l'amalgame, détestable, entre asile et immigration irrégulière, ensuite, parce que cette loi veut être un épouvantail dissuasif, qui n'aborde pas la seule vraie question : celle des moyens humains et financiers, renforcés lors du précédent quinquennat. Maîtriser l'immigration ? Vous savez, comme nous tous ici, que la maîtrise de l'immigration est d'abord une problématique européenne qui ne se réglera qu'au niveau européen. Le Président de la République ne dit pas autre chose. Comment la France seule pourrait-elle se prévaloir de maîtriser l'immigration, alors même qu'elle n'est que rarement le pays d'entrée en Europe ? La polémique récente avec nos voisins italiens a bien rappelé ce problème de l'inégalité européenne face au flux de migrants. Oui, notre continent subit depuis près de cinq ans la plus grande crise migratoire connue en Europe depuis les déplacements de populations consécutifs à la Seconde Guerre mondiale. Ce constat avait été fait dès l'été 2014 par le ministre de l'intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, qui fit alors une tournée d'Europe pour que des mesures soient prises. L'Europe a tardé avant d'adopter un mécanisme de répartition, de renforcer FRONTEX ou encore de créer des points d'accueil. Nous avons été fiers de défendre cette action de la France auprès de ses voisins. Le ministre d'État Gérard Collomb a mis en garde, ici même, et à juste titre, le 20 juin dernier dernier : « L'Europe peut se démanteler sur les problèmes migratoires. » Votre responsabilité n'est alors pas d'aggraver la situation avec une loi contestable et isolationniste, mais de faire vivre la solidarité européenne, madame la ministre. L'échec de la rencontre de Bruxelles de ce week-end a encore montré toute la difficulté de ce défi. Aujourd'hui, c'est n'est plus un défi, c'est une impasse. Alors, améliorer le droit d'asile, le deuxième grand thème de votre loi loi ? Comment pouvez-vous considérer que le droit d'asile sera amélioré en contraignant le délai de la demande et les conditions d'examen de cette dernière ? Vous ne réussirez avec vos mesures qu'à affaiblir l'accueil des demandeurs d'asile. La situation humanitaire de ces personnes s'aggravera de fait encore, puisque beaucoup ne pourront plus défendre leur demande dans de bonnes conditions. L'objectif d'accélérer l'examen des demandes est louable ; nous l'avons nous-mêmes porté lors du dernier quinquennat et vous l'aviez d'ailleurs soutenu à l'époque, avec Gérard Collomb. Et cet objectif a été rempli par la loi de 2015, qui n'est de pleine application que depuis trois ans. Pourquoi encore changer ces règles, sans évaluation de la précédente loi, et en intervenant cette fois sur les conditions même de la demande ? Et, là encore, il y a derrière cette problématique un sujet européen. La loi de 2015 est sans doute allée au bout de ce que nous pouvions faire en termes de pays d'accueil concernant l'asile. Le droit d'asile européen est à ce stade une pure fiction, laquelle se heurte aux égoïsmes qui sentent l'odeur du nationalisme exacerbé. Le dispositif de Dublin est mieux que rien, mais aussi peut-être pire que tout. Nous avons proposé, avec Jean-Yves Leconte, notre chef de file sur ce texte que je remercie, un amendement sur le sujet. Il a été rejeté. Encore une occasion manquée ... Troisième grand sujet, réussir l'intégration. Nous arrivons là au volet qui devait « équilibrer » votre projet de loi, en permettant l'intégration de ceux qui sont arrivés ces dernières années, alors que le flux commence à diminuer. Seulement, vous avez oublié un élément : quand il s'agit de principes fondamentaux de notre droit, il ne peut être question d'équilibre. On ne peut pas pondérer une remise en cause de nos valeurs et principes. Rien ne peut avoir suffisamment de poids pour équilibrer la balance quand, par ailleurs, vous en détraquez le mécanisme. Nous en sommes là, avec votre projet de loi. Nous prenons acte de certaines mesures, supprimées ou dénaturées par la droite sénatoriale. Mais jamais elles ne pèseront suffisamment pour que nous abandonnions les principes que nous défendons avec constance, en premier lieu desquels l'accueil digne et le droit d'asile. Alors, madame la ministre, nous ne comprenons pas le sens de votre loi, ou plutôt nous en avons bien compris la visée, le message. Cette loi n'est pas une loi de fermeté, c'est une loi de fermeture Vous faites écho, avec votre texte, à la tendance du repli et du court-termisme. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous : notre pays, par son histoire et par ce qu'il représente dans le monde, n'aura jamais l'image que vous cherchez à lui donner avec cette loi. C'est bien mal connaître les motivations des migrants et des réfugiés de penser qu'ils renonceront à venir en Europe ou en France du fait d'une simple loi. La conséquence de tout cela est simple : ils continueront à venir, mais ils seront moins bien accueillis et la situation humanitaire s'aggravera Vous aurez au moins réussi une chose avec ce texte, qui n'est qu'une loi d'affichage politique : à libérer les plus tristes passions anti-étrangers sur certaines travées parlementaires. Vous aurez permis la surenchère. La majorité sénatoriale- la droite de notre hémicycle -a embrayé, malgré sa faible mobilisation lors du débat, dans votre course à la fermeture du pays. Elle a encore aggravé les mesures contenues dans votre texte sur la rétention et le droit d'asile. Elle a aussi réduit les possibilités d'étude en France des étrangers, un bond de dix ans en arrière, indigne de notre pays et incohérent avec les objectifs d'excellence universitaire. Monsieur le rapporteur, vous et votre groupe avez porté dans ce débat des propositions que nous continuerons à combattre. Et ce que je disais au Gouvernement vaut aussi pour vous : vous ne réussirez pas à dissuader les migrants et à changer l'image de pays accueillant qu'est la France. France. Mes chers collègues, vous l'avez compris, nous aurions voté contre le texte sorti de l'Assemblée nationale. Nous voterons, avec encore plus de détermination, contre le texte modifié par la droite du Sénat. à l'amalgame entre asile, immigration et fraude, érigé en principe fondateur de ce texte, nous préférons résister aux peurs plutôt que les encourager nous préférons protéger les plus faibles plutôt que les rejeter ; nous préférons intégrer sur la base des valeurs de la République plutôt que précariser. En conclusion, je voudrais vous inviter, en ce jour anniversaire du chantre de la fraternité universelle,

la question migratoire, sujet sensible pour les Français s'il en est, est devenue un enjeu de souveraineté nationale et de cohésion sociale. Illustration Illustration de cette importance, nos débats ont été passionnés, parfois difficiles, mais à la hauteur d'un enjeu fort pour nos concitoyens. Un enjeu fort, car nos concitoyens constatent que le phénomène n'est toujours pas enrayé. Alors que les demandes d'asile refluent partout en Europe, elles augmentent en France. Comme l'a affirmé le Président de la République dimanche dernier, la France est le deuxième pays d'accueil en Europe pour cette année. Quelques chiffres pays a délivré 262 000 titres de séjour en 2017 ; plus de 300 000 étrangers en situation irrégulière sont inscrits à l'aide médicale de l'État. Quant au nombre de demandeurs d'asile, il a lui aussi franchi un record, avec plus de 100 000 demandes déposées l'an dernier. selon la Cour des comptes, 96 % des déboutés du droit d'asile restent dans notre pays. À la lecture de ces chiffres, vous comprenez, madame la ministre, mes chers collègues, que la situation est intenable. Elle est d'autant plus tendue que nos procédures de traitement et les dispositifs d'hébergement sont d'ores et déjà saturés, particulièrement en Île-de-France et dans le Pas-de-Calais, où se constituent des campements illégaux, au détriment de tous, surtout des riverains et des pouvoirs publics. Quant à la question de l'intégration des étrangers dans notre pays, leur insertion linguistique, économique et sociale est particulièrement insuffisante en comparaison de belles réussites chez nos partenaires, notamment chez nos Ce projet de loi ne peut laisser insensible, puisqu'il tente d'apporter une réponse à un défi immense et complexe. Aussi, nul ne peut prétendre détenir la vérité absolue, nul ne peut prétendre au « monopole du coeur », quelles que soient les responsabilités et les sensibilités politiques de chacun d'entre nous. En effet, mes chers collègues, on peut constater une continuité politique assez nette sur le sujet de l'immigration entre tous les gouvernements depuis plus de vingt ans. Cette continuité est celle de la recherche d'un équilibre entre l'immigration, l'intégration et le droit d'asile. C'est aussi celle d'une cohérence de ces trois enjeux majeurs, qui sont encore une fois abordés ici dans un seul et même texte. Le gouvernement actuel est resté dans la droite ligne de la tradition française, l'esprit de ce texte était donc le bon. Néanmoins, il pouvait être amélioré, en faisant preuve d'un pragmatisme qui a guidé la commission des lois de notre assemblée. En effet, si notre commission est allée assez loin sur certains sujets, elle a également fait oeuvre d'amélioration et de réalisme sur d'autres. Nos débats et les ajustements apportés en séance ont permis de prendre en compte les préoccupations de certains de nos collègues et des ajouts du Gouvernement. Un certain nombre de dispositions ont ainsi été apportées. Elles vous aideront à donner des réponses cohérentes à des difficultés techniques. C'est pourquoi nous appelons de nos voeux la construction d'une réponse globale et stratégique à ces défis qui ne feront que s'accroître et s'intensifier. Pour apporter une réponse globale à cette question, il faut deux choses : de la volonté politique et des moyens financiers. De la volonté, il vous en faudra, madame la ministre, pour contrôler l'application de cette loi et faire enfin respecter l'intégralité des dispositions de notre droit. Il faudra d'ailleurs plus que des mesures techniques pour régler la question, nous devrons avoir une grande stratégie. Dans un contexte différent certes, mais confronté à la même urgence, le général de Gaulle appelait en mars 1945 à un grand plan national « afin afin d'introduire au cours des prochaines années, avec méthode et intelligence, des éléments d'immigration dans la collectivité française ». Inspirons-nous de cette démarche, madame la ministre, afin de proposer une vision politique du problème. En ce qui concerne le financement, le compte n'y est pas, tant s'en faut. Nous aurons beau adopter les textes les plus complets du monde, tant que nos forces de l'ordre, nos magistrats, magistrats, nos interprètes, bref tant que tous nos fonctionnaires de l'asile continueront à oeuvrer dans des conditions déplorables, nous ne réglerons rien. À titre d'exemple, la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, avec plus de 53 000 demandes d'entrée en 2017, a connu une progression du nombre de dossiers de 34 % par rapport à 2016. Plus d'un tiers d'augmentation ! Ces chiffres sont impressionnants et nous devrons nous en souvenir lors des discussions sur le budget pour 2019. Enfin, c'est bien au niveau européen que doit être portée cette question. Nous espérons que les chefs d'État et de gouvernement réunis en Conseil européen cette semaine parviendront à un accord équilibré sur la réforme du régime d'asile européen. Le sommet de dimanche dernier n'est malheureusement pas de bon augure : l'Europe apparaît divisée et prisonnière des agendas politiques des uns et des autres. La France devra défendre une approche conforme à sa tradition de responsabilité et d'humanisme. Elle devra s'efforcer d'obtenir un consensus sur ce sujet qui divise l'Europe. Elle devra redonner corps à la promesse européenne de sécurité, de prospérité et de responsabilité. Si nous échouons, en Europe, si vous échouez, madame la ministre, tous nos débats n'auront servi à rien. Cet énième texte sur l'immigration, malgré votre bonne volonté, restera une coquille vide.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, par le passé, l'immigration conduisait à l'assimilation. Aujourd'hui, l'immigration conduit au communautarisme et les flux migratoires sont une menace pour l'avenir. Pour que la France reste la France, il est urgent de reprendre notre destin en main. Je n'accepte ni le fatalisme de ceux qui prétendent qu'on ne peut rien faire ni, pire encore, l'irresponsabilité de ceux qui soutiennent cette invasion migratoire. Certains pays européens ont fait preuve de détermination, et ils sont parvenus à endiguer ces flux migratoires. C'est le cas de la Pologne et de la Hongrie et, depuis peu, de l'Autriche et de l'Italie. Tout comme eux, nous devons fermer nos frontières, supprimer les aides sociales qui servent d'appel d'air, expulser les clandestins en situation irrégulière, expulser aussi tout étranger qui commet un crime ou un délit sur notre sol. Enfin, il faut mettre un terme au laxisme à l'égard du communautarisme et de l'extrémisme musulmans. Comme le reconnaît lui-même l'actuel ministre de l'intérieur, nos aides sociales sont une véritable pompe aspirante, car les migrants choisissent systématiquement les pays où ils profitent du maximum d'aides sociales. En raison des difficultés économiques et des restrictions budgétaires, nous devrions d'abord régler les problèmes de nos concitoyens avant de nous occuper de ceux des autres. Ainsi, le 13 octobre 2015 à la tribune du Sénat, j'avais déjà dit combien il est scandaleux que certaines veuves d'agriculteur ou de petit commerçant ne perçoivent que 300 euros par mois, alors que chaque migrant nous coûte au total plus de 1 000 euros par mois. C'est lors de cette même intervention, j'avais dit que l'immigration d'aujourd'hui, c'est le vivier de recrutement du terrorisme de demain. Tous les bien-pensants avaient alors hurlé en criant au scandale. Or, trois semaines après, les attentats du Bataclan m'ont donné raison. Amalgame ! Deux terroristes venaient d'entrer en France en tant que demandeurs d'asile. Plus récemment, il y a un mois, on a découvert que nous hébergions un bourreau de l'État islamique recherché par toutes les polices. Or, non seulement il avait été régularisé au titre de l'asile des migrants, mais en plus il percevait les aides financières de l'État Quand on énumère ces faits, les tenants de la pensée unique crient à l'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame, c'est seulement la terrible réalité. Cela doit cesser. La France doit rester la France. Merci seuls quelques responsables politiques ont eu le courage de le dire. À son tour, M. Wauquiez a diffusé un tract : « Pour que la France reste la France

nous laissons dix secondes à M. Masson. S'il croit ce qu'il dit, il doit accepter de travailler avec ceux qui, bien avant lui, ont toujours été clairs sur ce sujet. À défaut, lors des prochaines échéances électorales, les Français sauront faire la différence

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je crois que nous partageons tous dans les grandes lignes le constat dressé par notre rapporteur concernant le fonctionnement actuel du système d'accueil et d'intégration des étrangers sur notre territoire : la saturation de nos capacités d'hébergement d'urgence, qui menace la dignité des demandeurs d'asile les difficultés de l'État à faire respecter les décisions de refus d'admission à l'asile et au séjour, et les décisions d'éloignement qui en découlent l'insuffisance des moyens consacrés à l'intégration des personnes étrangères en situation régulière sur notre territoire. Il est donc regrettable que nous ne soyons pas parvenus à dépasser nos clivages politiques, afin de nous livrer à une évaluation scrupuleuse des dispositifs actuels et de leurs limites. J'avais déjà évoqué, lors de la discussion générale, la position de notre groupe sur le sujet : la dimension prospective est excessivement laissée de côté. Peu de choses sur les outre-mer, qui pour beaucoup sont perçus comme une porte d'entrée vers la France et l'Europe. Rien sur la remise à plat des instruments de développement français. La proposition de notre collègue M. Thani Mohamed Soilihi et les échanges qui en ont découlé ont révélé également la difficulté de légiférer sur l'admission au séjour sans discuter à la fois des conditions d'attribution de de la nationalité française. Une approche globale nous a manqué. Sans anticiper les discussions en cours sur l'évolution du système de Dublin, le texte se borne, pour l'essentiel, à modifier de nouveau les aspects procéduraux des demandes d'asile et d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière. Malgré quelques modifications progressistes aux marges du texte, venues de la gauche de l'hémicycle, le rééquilibrage proposé par notre rapporteur ne nous convient pas tout à fait, dès lors qu'il déplace le curseur de la fermeté à l'égard des étrangers en attente de décision ou en situation irrégulière, sans adapter celui de la protection de leurs droits et libertés fondamentales. Cet équilibre est pourtant précieux. Comme l'écrivait Blaise Pascal, « la justice sans la force est impuissante, mais la force sans justice est tyrannique ». Mes chers collègues, je connais l'attachement de notre Haute Assemblée à la protection des droits et des libertés fondamentales. Quel peut être le sens d'un État de droit qui protégerait moins les individus en situation de vulnérabilité, et mieux les individus qui connaissent leurs droits et entendent les exercer pleinement ? C'est pourtant le sens de ce texte, qui prévoit de renforcer les dispositions procédurales dérogatoires pour les administrés étrangers, que ce soit le recours à des audiences par l'intermédiaire de captations vidéo, l'inflexion des règles relatives à la notification, l'extension des cas de recours devant un juge unique ou encore, dans certains cas, la suppression de l'effet suspensif du recours.

Si nous attendons des étrangers présents sur notre sol qu'ils se conforment aux lois de la République, il nous revient de nous assurer qu'ils puissent accéder à nos juges dans des conditions conformes à notre héritage juridique. En effet, dans bien des contentieux, l'accès au juge a pour fonction non pas seulement de rendre justice, mais également de faire entendre justice auprès des publics les moins informés de nos règles de droit. Sur ces sujets, nous devons veiller à ne pas appauvrir le débat en le réduisant à la seule question de la conformité à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou aux textes européens qui nous lient. Nous savons dans quel contexte ont été adoptés les règlements de Dublin. Il fallait obtenir une rédaction offrant des marges de manoeuvre, afin qu'elle puisse convenir à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, dans lesquels les garanties offertes aux justiciables diffèrent sensiblement des nôtres. Je crois qu'il revient au législateur de prendre une position plus claire, plutôt que de se cacher derrière les latitudes offertes par d'autres textes, d'autres autorités, et d'assumer ses choix. C'est pourquoi, par souci de fidélité à nos valeurs séculaires, mes collègues du groupe du RDSE et moi-même avons exprimé notre opposition, quand nos valeurs et notre conception de la justice étaient mises à mal. Ce fut notamment le cas à propos de la faculté de retenir en centre de rétention administrative des mineurs accompagnés de leurs parents, plutôt que de les soumettre à assignation à résidence.

ou encore un encadrement plus important de l'accès aux fonctions d'interprète. Mais même ce second point est considérablement atténué par la possibilité de maintenir l'interprète à distance du requérant étranger lors d'une vidéo-audience, qui reste dans le texte adopté par le Sénat. Après les longs débats que nous avons eus sur ce projet de loi, débats qui, sur certains sujets, auraient mérité d'être plus longs encore, les membres du groupe du RDSE voteront contre le texte proposé par la droite sénatoriale.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous arrivons au terme de la semaine d'étude de ce texte.

des vingt-neuf textes votés depuis 1980 et des seize textes majeurs qui ont concerné l'asile et l'immigration.

c'est très clair ; sur la procédure d'asile, nous avions des éléments à discuter ; sur l'immigration irrégulière, il reste, malgré quelques avancées, faible.

Dans ces conditions, le groupe Les Républicains a décidé de reconstruire ce texte, de le réécrire et de lui donner un peu de sens, ... Très bien ! ... sur le fondement d'une stratégie politique claire, que je vais rappeler. rappeler. Tout d'abord, nous sommes favorables à une politique d'intégration digne de ce nom. Nous préférons recevoir moins, mais recevoir beaucoup mieux que ce que nous faisons depuis des années. nous avons souhaité que, en matière d'asile, les procédures et les efforts entrepris depuis plusieurs années se poursuivent, afin que la procédure soit la plus courte possible la plus courte possible et que la protection que nous devons à ceux qui doivent être protégés, et que la France accorde, soit offerte dans des délais rapides. Néanmoins, cette procédure ne doit pas être pour les réseaux de passeurs le moyen absolu d'une immigration irrégulière incontrôlée.

Nous avons fait évoluer le texte. Il faut faire sortir de la tête de nos concitoyens que tous les migrants, tous les étrangers, sont des réfugiés.

dire les choses, c'est essayer de se donner la chance de trouver des solutions ; ce débat est donc absolument nécessaire. Nous avons tenté, bien sûr, de trouver des solutions pour Mayotte à la faveur d'un amendement déposé par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, nous avons adapté une partie du droit du sol. Nous avons demandé que le Gouvernement puisse conditionner l'accord de visas de long séjour

Nous avons d'abord réglé le problème des mineurs, en interdisant très clairement leur placement en rétention. Nous n'avons pas accepté qu'une famille avec enfants puisse être placée en rétention durant plus de cinq jours Je me permets de rappeler à tous ceux qui n'ont pas voté pour l'amendement

à condition d'en définir les critères et les conditions. C'est ce que nous avons essayé de faire. Très bien ! En outre, une politique migratoire doit s'inscrire dans le temps. Nous avons besoin de ce texte, tel qu'il sortira de la Haute Assemblée, pour l'inscrire dans la durée.

considérez simplement que la réforme du régime dit « Dublin » a débuté en 2014 et que nous sommes en 2018 ! Les choses n'avancent pas ... Je veux saluer le travail de la diplomatie parlementaire. Cette semaine, le président du Sénat est allé, avec le président de l'Assemblée nationale, au Maroc. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ils indiquent très clairement leur volonté de lutter contre l'immigration irrégulière et de s'inscrire dans des accords de coopération étroits, étroits, bilatéraux ou multilatéraux. Cela doit être salué et cela montre l'utilité de ces coopérations parlementaires. Enfin, je veux remercier l'ensemble des

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre échange de cet après-midi conclut un débat intense, complet, prolongé, auquel beaucoup ont participé et qui a permis d'aboutir à des clarifications.

renforcer l'intégration, en particulier en maintenant ouverts les mécanismes de réunion des familles, et, oui, fournir des moyens effectifs de reconduire à la frontière les personnes dont le droit au séjour n'est pas reconnu par notre loi. en effet que le choix politique d'améliorer le contrôle du maintien sur le territoire français constitue une responsabilité régalienne que notre pays doit pleinement assumer, en tenant compte des équilibres sociaux qui sont associés à l'effort d'intégration, mais aussi des limites de la capacité d'intégration. Bien sûr, nous avons tous le souhait que cela se réalise dans la coopération européenne, mais j'y insiste, il faut parler de coopération, car il s'agit d'une compétence souveraine de chacun des États.

Donc, ne pensons pas que nous pouvons nous libérer de nos propres responsabilités nationales en croyant à un accord européen complet, malheureusement loin de notre portée. le projet de loi a donné lieu à beaucoup de points d'accord sur des mesures ponctuelles, et à des améliorations- j'espère, madame la ministre, que le Gouvernement en tiendra compte dans la suite du débat, dans le respect du bicamérisme. Je veux à cet égard remercier François-Noël Buffet et saluer son travail comme rapporteur ; il a fait un travail très important dans un état d'esprit de rapprochement et de compréhension- je parle du rapporteur et non de l'orateur qui m'a précédé

J'en cite simplement quelques-uns : le remplacement de l'aide médicale d'État par un système inconnu à ce jour, et qui rappelle d'ailleurs quelques débats anciens sur la définition des maladies graves ; ... C'est

l'exclusion de toute aide au transport imposée aux autorités locales ; ou encore la limitation excessive du droit de la réunion des familles.

de présentation, de démonstration, qui ne peuvent pas avoir d'effet pratique. C'est ce qui conduit le groupe La République En Marche à ne pas donner son accord au projet de loi ainsi déformé, et à émettre un vote négatif

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est une toile de fond bien sinistre qui s'est déployée lors de la discussion de ce texte au Sénat. de la journée mondiale des réfugiés, a publié un cahier d'une soixantaine de pages contenant la liste de 34 361 migrants et réfugiés morts depuis 1993 en essayant de pénétrer la « forteresse Europe D'outre-Atlantique, nous sont parvenues des images effarantes de camps de rétention, où des enfants séparés de leurs parents sont enfermés en cage, nourrissons compris. compris. En Méditerranée, après avoir parcouru 1 500 kilomètres et être passés à 7 kilomètres des côtes françaises, 629 migrants, ballottés sur la « grande bleue », ont finalement trouvé refuge à Valence, en Espagne, la semaine dernière.

-ou dans les pays ne les accueillant pas- position franco-allemande. En 2015, la question posée à l'échelon européen était : comment répartit-on les réfugiés ? Aujourd'hui, avec pour boussole la position de gouvernements conservateurs alliés aux néo-fascistes, on se demande : comment les empêche-t-on d'arriver ? Le Président Macron fait le grand écart : à Bruxelles, il sermonne les États anti-migrants et, en France, il bloque les ports. C'est l'hôpital qui se fiche de la charité En réalité, le pays des droits de l'homme s'échappe et tend à se refermer sur lui-même dans un double objectif : montrer aux migrants qu'il ne faut surtout pas demander l'asile en France rassurer les électeurs ou sympathisants d'extrême droite, puisque les conditions sont créées pour bafouer le droit d'asile et mettre à mal l'accueil de migrants à tout autre titre. un objectif légèrement différent, mais en tout cas avec les mêmes finalités, la majorité sénatoriale a fait adopter l'instauration de quotas qu'évaluerait chaque année le Parlement, sans se soucier réellement des causes profondes qui conduisent à ce monde de migrations et de réfugiés. A été actée la disparition de l'aide médicale d'État, remplacée par un dispositif d'urgence, au moment même où Médecins du monde et le centre Primo-Levi ont publié un rapport sur les traumatismes dont souffrent les exilés, aggravés par l'errance qui leur est infligée en France- tentatives de suicide, automutilations, décomposition, addictions et développement de troubles psychiatriques. Le délit de solidarité, quelque peu assoupli par l'Assemblée nationale, qui avait exempté de poursuites les personnes qui apportent une aide à la circulation aux migrants, a été rétabli dans sa version existante, continuant ainsi à criminaliser ceux d'entre nous qui apportent en toute fraternité aide et soutien aux exilés. Un amendement adopté est, selon nous, particulièrement grave : il ouvre une brèche dans le droit du sol à Mayotte. Nous espérons que la commission mixte paritaire échouera précisément sur ce point et qu'un projet de loi en bonne et due forme permettra la tenue d'un vrai débat et la présentation par le Gouvernement de son ambition pour résoudre la crise qui sévit dans ce département français, sans remettre en cause notre droit de la nationalité. Enfin, en matière de rétention, derrière sa cape de « défenseur des libertés », la commission des lois du Sénat avait introduit plusieurs mesures « d'assouplissement » revenant sur la disposition phare de Gérard Collomb, qui portait à 90 jours la durée maximale de rétention, et rétablissant la durée de la première phase de rétention administrative a été rallongée à cinq jours, contre quarante-huit heures actuellement. En outre, a été gravée dans la loi une durée maximale d'enfermement pour les mineurs avec leur famille de cinq jours, qui légalise de fait l'enfermement des mineurs avec leur famille sur notre sol. En résumé, ce projet de loi et son examen au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, n'ont eu de cesse de déshumaniser le sujet dont il est question, ...

très révolutionnaire de notre politique migratoire ; il s'agissait simplement d'améliorer les conditions de vie et d'accueil des personnes, en respectant l'intérêt supérieur de l'enfant, en veillant notamment aux droits fondamentaux- un toit, la santé et les besoins alimentaires, ainsi que, éventuellement, les mêmes droits de recours que pour tout justiciable, et un accès facilité au travail. En outre, ces amendements tendaient à garantir le respect des principes fondamentaux auxquels notre pays a souscrit dans sa Constitution et dans ses engagements internationaux. Dans une Europe en proie à la montée des nationalismes, la France doit prendre ses responsabilités et réaffirmer les valeurs qu'elle a toujours portées, celles qui fondent notre République. La Banque

ce projet de loi auquel nous demeurons opposés ne propose aucune issue à ce défi humanitaire.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'histoire s'est accélérée en une semaine. Depuis mardi dernier, a témoigné d'un malaise, il ne faut pas le cacher. Il a témoigné de notre interrogation face aux migrations, ainsi que face à une remise en cause de la construction européenne, mais aussi des modes de régulation pensés par les Européens depuis longtemps, tant pour eux que pour la scène internationale. Quand l'histoire s'accélère, elle exige la clarification,

par l'Europe ; vous le savez, c'est notre première idée directrice : plus d'Europe, une Europe plus forte et plus aboutie. La solution en matière d'asile et d'immigration ne sera pas franco-française, elle sera européenne. Que Que l'on parle de FRONTEX, de la révision du règlement de Dublin, des centres fermés, de zones d'attentes de centres d'accueil dans les pays d'origine, de la définition du droit d'asile- nous pourrions continuer la liste -, nous sommes interdépendants. Exprimée autrement, notre conviction est que la souveraineté française trouve aujourd'hui sa pleine expression, sa pleine mise en oeuvre, dans une souveraineté partagée. il y aura, chers collègues, une solution européenne ; nous vous faisons confiance, madame la ministre, nous faisons confiance au Gouvernement et nous faisons bien entendu confiance au Président de la République- chacun sait combien il est moteur sur

probablement inaccessible à l'heure actuelle. La deuxième solution, prévue par les traités européens, résiderait dans une coopération renforcée, la fameuse « Europe à plusieurs vitesses » avec un premier noyau qui ferait le choix d'aller plus loin, en rappelant que le droit d'asile n'est pas soumis à règle de l'unanimité par le traité de l'Union européenne.

chers collègues, quelle que soit la solution, celle-ci aura une traduction législative, ce qui me conduit à la deuxième idée directrice du groupe Union Centriste, qui consiste à analyser le texte qui nous est soumis comme un texte de transition,

Notre pays a réagi à des crises successives, notamment en 2015. Le terme de « crise » n'est d'ailleurs plus adapté ; nous affrontons un problème de long terme, des migrations qui ont changé de nature et qui s'inscrivent dans la durée. La réponse aux migrations sera la responsabilité de toute une génération. Nous voterons le texte proposé, même si notre ligne de crête « ni angélisme ni surenchère » a connu quelques défaillances. Sans entrer dans le détail technique,

Ne vous trompez donc pas sur le décompte des voix qui sera annoncé tout à l'heure. Chers collègues partenaires de la majorité sénatoriale, le groupe Union Centriste n'adopte pas et n'adoptera pas un contre-projet à celui du Gouvernement. Très bien ! Nous adoptons une base de négociation pour un rapprochement souhaité avec l'Assemblée nationale, dans le respect de chacun, sur un sujet, à notre sens, d'unité nationale ! Chers collègues ! Chers collègues communistes ou socialistes, si nous n'avons pas soutenu vos salves d'amendements, nous reconnaissons que vous nous avez posé une très bonne question quel point l'adoption de mesures plus restrictives est-elle de nature à redonner confiance à nos concitoyens et à éviter la progression des populismes ? Eh oui ! Où est la limite qui ferait de nous les otages d'une surenchère permanente ? Notre réponse, en particulier sur le droit d'asile, est l'État de droit- non pas la morale ni des valeurs non définies, mais bien des règles de droit précisées au cours des décennies par nos Constitutions successives, par des principes fondamentaux à valeur constitutionnelle, par les règles conventionnelles. C'est la définition même de l'État de droit et notre meilleure garantie face aux peurs et à l'émotion. Je vous renouvelle, madame la ministre, notre confiance pour nous aider

saluer plus particulièrement M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur, qui ont contribué à un débat fourni. remercier les vice-présidents qui se sont succédé au plateau : ils ont tous contribué au bon déroulement des travaux parlementaires.

La diplomatie n'est pas toujours facile, mais elle est conduite avec beaucoup de volontarisme de la part du Président de la République, du Premier ministre et du ministre d'État, ministre de l'intérieur. J'en profite pour remercier

depuis trop longtemps, ce que l'État ne rembourse pas aux départements qui versent les allocations de solidarité pour le compte de la Nation. Depuis 2012, de négociations en négociations avec les gouvernements successifs, on achoppe sur le financement des politiques de solidarité.

qui a été interprété comme un chantage et un autoritarisme déplacé. La France, pour se redresser, a besoin de tous, de l'État comme des collectivités locales, chacun devant consentir sa propre part d'efforts. Les relations à construire entre l'État et les collectivités doivent reposer sur une confiance réciproque et sur une vraie concertation.

vous répondre, d'évoquer la question de la nature des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, plus particulièrement les départements, puisque c'est sur la situation de ces derniers que vous appelez l'attention du Gouvernement. Depuis longtemps- vous l'avez dit -, depuis bien avant la nomination de ce gouvernement, sous de très nombreuses majorités successives, les relations financières entre l'État et les départements sont compliquées. le sont en raison du dynamisme de la dépense sociale. Le dynamisme des dépenses sociales dites « AIS » est tel que les départements doivent consentir un effort considérable pour y faire face. De la même façon, depuis quelques années,

Conscients de ces difficultés, les gouvernements successifs ont, année après année, décidé d'accorder des fonds d'urgence aux départements.

S'agissant des MNA, nous avons formulé une proposition fondée sur une reprise en main par l'État d'un certain nombre d'éléments de responsabilité avant le moment où un mineur est déclaré- ou non -mineur non accompagné.

Premier ministre, je souhaite que tout soit mis en oeuvre pour mettre fin aux incompréhensions entre l'État et les collectivités, en particulier les départements. Nous

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités Madame la ministre, vous avez engagé une réflexion sur les pensions de réversion, et, depuis une semaine, vous vous êtes expliquée sur ce sujet. Vous avez notamment affirmé que vous ne toucherez pas aux pensions déjà versées et que l'acquis serait maintenu. Malgré tout, sachez que l'ouverture de ce débat suscite de nombreuses inquiétudes. Vous le savez, la pension de réversion concerne à 90 % des femmes. Il est vrai que l'espérance de vie est plus importante pour une femme que pour un homme, comme nous le savons toutes et tous ici. il s'agit aussi, par cette pension de réversion, d'améliorer la situation de nombre de femmes qui ont connu des carrières incomplètes ou des différences de salaire importantes avec les hommes. Au travers de cette question, je souhaite que vous nous apportiez des précisions sur les critères que vous pensez retenir pour cette éventuelle réforme et sur la manière dont vous allez prendre en compte, dans vos calculs, les nouvelles formes de familles, comme les couples pacsés ou les familles recomposées. Madame Madame la ministre, après la hausse de la CSG, avec l'annonce de cette réforme des pensions de réversion, les retraités sont une fois de plus pointés du doigt et se retrouvent dans l'incertitude. Ainsi, plus tôt vous annoncerez vos orientations, plus tôt vous pourrez rassurer,

le Gouvernement a eu l'occasion d'indiquer que le programme de travail que nous nous fixions comporterait, avant septembre 2017, une transformation du droit du travail- les ordonnances ont été adoptées depuis

et parce que la diversité des régimes applicables et la sensibilité de nos concitoyens à l'avenir de leur pension sont telles que la précipitation et l'urgence seraient évidemment contre-productives. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé, avec Mme la ministre des solidarités et de la santé, à la nomination d'un haut-commissaire, dont la mission

-à cette réflexion et à cette consultation sur ce que sera, demain, notre système de retraite. Pour cela, j'ai fixé quelques objectifs très simples : la préservation d'un système de retraite par répartition,

les bénéficiaires de ces pensions se trouvent dans des situations incroyablement diverses. Comme tous les aspects du système de retraite, nous devons poser sur la table la question les pensions de réversion. Il ne s'agit évidemment pas de les faire disparaître. pas à nous faire peur ! Il n'est absolument pas question de revenir sur cet élément indispensable en matière de solidarité et de complément de revenu pour des femmes qui, bien souvent, ont participé à une activité de production ou ont dû interrompre leur activité pour élever leurs enfants.

verra un très beau débat public et un très beau débat parlementaire. Il nous faudra faire en sorte de sauver notre système de pensions durablement et, peut-être, en profiter pour prendre en compte des questions relatives à la dépendance, un sujet qui n'a pas fini être devant nous. La parole

Je ne vous cacherai pas, madame la ministre, l'inquiétude qui remonte de la population sur le sujet des pensions de réversion. Certes, me direz-vous, des démentis ont été apportés, y compris par vous-même, mais le mal est fait : la rumeur, qui est le plus vieux média du monde

Cette volonté d'harmonisation est au coeur du projet de réforme des retraites en préparation, qui a pour objectif l'instauration d'un régime universel en établissant ce qui relève de l'ordre de la redistribution et de l'ordre de la solidarité.

C'est au prix de certaines clarifications, dès le départ, que le débat pourra s'engager d'une façon sereine, car je ne doute pas que votre volonté n'est pas de réformer pour réformer, ni même de réformer pour réduire les droits ou pour les niveler par le bas,

concerne la construction d'un système redistributif et solidaire. Il s'agit de poser la question des droits non contributifs liés à la maternité, au chômage, à l'assurance maladie, Le troisième bloc a trait aux évolutions de la société et donc aux droits familiaux. C'est dans ce cadre que se pose la question des pensions de réversion, raison pour laquelle cette thématique a émergé au cours de la concertation et dans les contributions sur le site internet qui permet aux citoyens de s'exprimer.

solidarités et de la santé. Madame la ministre, vous étiez entendue ce matin par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'égal accès aux soins,

et alertent sur une mise en danger de la vie d'autrui, faute de moyens suffisants et d'une organisation efficiente de l'offre de soins. Les services d'urgences sont les plus touchés et la situation devrait même s'aggraver : d'après une étude de l'agence régionale de santé Île-de-France, au cours des deux

qui apparaît comme une solution dégradée face à la pénurie de praticiens. Dans mon département de Meurthe-et-Moselle, la maternité de l'hôpital de Mont-Saint-Martin est menacée de fermeture en raison d'un nombre considéré comme excessif de médecins remplaçants, qui pallient pourtant la pénurie à laquelle nous sommes tout particulièrement confrontés. Cette maternité, avec ses 670 naissances chaque année, a toute sa place sur un territoire transfrontalier en pleine renaissance post-industrielle, où le préfet de région s'est vu tout récemment confier une mission de prospective de dynamisation par le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard. Madame la ministre, vous ne portez pas la responsabilité du manque de réformes de vos prédécesseurs. Vous avez eu le courage d'annoncer une refonte en profondeur du système de santé pouvez-vous nous dire quelle place vous comptez accorder aux hôpitaux de proximité ? Êtes-vous en mesure de rassurer les habitants de mon territoire sur le maintien de la maternité contribuant à l'attractivité de l'hôpital et à l'attractivité médicale de tout un territoire ?

médecins urgentistes ont annoncé leur démission pour le 3 juillet prochain. Un ras-le-bol qui couvait depuis longtemps au CHAR, secoué de crises multiples, comme j'ai pu le constater en avril dernier, lors de la visite de la mission des affaires sociales à laquelle je participais : bâtiment vétuste, nombre insuffisant de lits, manque de généralistes et de spécialistes, difficultés à fidéliser les professionnels de santé, médecine libérale défaillante ... En Guyane comme partout, les problèmes rencontrés aux urgences sont la résultante du dysfonctionnement du système de santé, ce que j'avais souligné, en juillet 2017, dans le rapport d'information de la commission des affaires sociales avec mes collègues Catherine Génisson et René-Paul Savary. Madame la ministre, pourriez-vous nous dire quelles mesures d'urgence vous comptez prendre pour combler le manque de praticiens à Cayenne, comme dans toute la Guyane et dans les autres départements ultramarins, qui vivent de manière plus aigüe la crise de notre système de santé ? Et pourquoi, avant d'agir, attendre des actions si lourdes de conséquences ici, la démission de praticiens, à Sotteville-lès-Rouen la grève de la faim à l'hôpital psychiatrique du Rouvray ou encore, dans la Nièvre, la démission de

favorable à la modernisation du centre hospitalier. Eu égard à la dégradation financière de l'établissement, une délégation de 40 millions d'euros, conformément aux accords de Guyane du 21 avril 2017, va être

chaque médecin est reçu chaque fois qu'il le demande, et nous faisons en sorte que l'ARS rencontre les médecins de ville pour leur suggérer de participer à la régulation des soins d'urgence.

de garde. Nous avons créé cent postes d'assistants spécialistes pour les DOM, mesure dont bénéficiera la Guyane dès cette année. Enfin, une nouvelle séquence de négociation est programmée aujourd'hui. Nous mettons tout en oeuvre pour qu'elle se termine par un projet d'accord final. Je terminerai en soulignant qu'une mission d'audit a été confiée au professeur Pierre Carli, président du Conseil national de l'urgence hospitalière, que tout le monde connaît. Elle aura lieu du 7 au 9 juillet prochain, pour évaluer la situation particulière des urgences de Cayenne. Des décisions seront prises ! Vous constatez notre mobilisation pleine et entière pour redresser cette situation dégradée. La parole

et pris possession de la stalle en la basilique Saint-Jean-de-Latran. Ce faisant, il s'inscrit dans les pas d'Henri IV, qui avait inauguré cette pratique en 1604, avant que la Révolution ne la fasse tomber en désuétude jusqu'en 1957. Il ne s'agit aucunement d'une obligation institutionnelle, puisque l'article 1 de notre Constitution se borne à rappeler que la France est une République laïque, qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion et qu'elle respecte toutes les croyances, tandis que l'article 2 de la loi de 1905 énonce que la République ne reconnaît aucun culte. Il ne s'agit pas non plus d'une coutume, puisque, dans la féconde histoire de notre république, seuls cinq présidents ont pris possession de ce titre- Georges Pompidou, François Mitterrand et François Hollande s'en sont tous les trois abstenus, ce qui ne les a pas empêchés d'avoir des relations diplomatiques constructives avec le Vatican. Il s'agit plutôt d'un énième dévoiement de la laïcité, au profit d'un oecuménisme communautariste qui affaiblit notre république.

Alors que votre majorité à l'Assemblée nationale se fissure une nouvelle fois à cause de l'opposition de certains de vos députés au souhait du Gouvernement d'exempter les « associations à but cultuel » de l'obligation de déclarer leurs actions de auprès des décideurs publics, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous expliquer le sens de cette visite, au moment où les fondements de notre république laïque sont affaiblis par les revendications identitaires et communautaristes

sur la laïcité, le Président de la République et les membres du Gouvernement n'ont jamais changé de ligne, celle d'un attachement profond à la loi de 1905,

doit pouvoir exercer son culte dans de bonnes conditions, ou alors ne pas croire, ce qui est une autre liberté. La visite d'État de ce jour

sur plusieurs thèmes, notamment l'émigration, dont nous avons beaucoup parlé, ici même, ces jours derniers, la lutte contre le dérèglement climatique, l'aide au développement, la situation des chrétiens d'Orient, mais aussi la protection des minorités. Je tiens également à préciser que le titre de chanoine du Latran, dont le président prendra officiellement possession, est un titre laïque, qui n'a aucune dimension spirituelle, mais possède uniquement une signification honorifique et historique. C'est une distinction, vous l'avez souligné, qui revient automatiquement au chef de l'État français depuis Henri IV. Pour être très précis historiquement, tous les Présidents de la République l'ont été,

qui pourrait bien déterminer l'avenir de la zone euro. Tout d'abord, elle a permis d'acter un accord sur la dette grecque et de rendre aux Grecs leur autonomie financière. Après presque une décennie de sacrifices, c'est un grand moment pour la Grèce, c'est un grand moment pour la France, qui s'est toujours tenue à ses côtés, et c'est un grand moment pour la zone euro, qui montre qu'elle est enfin capable de sortir de la crise. Ensuite, cette réunion a permis de présenter le programme de réforme de la zone euro, défini par Emmanuel Macron et Angela Merkel à Meseberg, la semaine dernière. Ce projet est équilibré il associe l'idée française d'un budget commun de la zone euro et la volonté allemande de créer un véritable Fonds monétaire européen. Il associe donc à égalité rigueur budgétaire et nécessité d'investir dans l'avenir.

Madame la secrétaire d'État, les questions que nous nous posons ne sont pas seulement techniques ; elles sont aussi politiques. La zone euro apparaît plus divisée que jamais. Votre homologue néerlandais a pris la tête d'une fronde de douze pays opposés au projet franco-allemand. Au sein même de la majorité d'Angela Merkel, plusieurs poids lourds s'opposent à ce que les Allemands payent pour les autres. La Chancelière est affaiblie, l'unité de l'Eurogroupe est rompue. La France apparaît bien seule pour porter une ambition européenne forte et crédible. Dans ce contexte, madame la secrétaire comment comptez-vous convaincre nos partenaires d'avancer avec nous pour réformer la zone euro et construire une union économique et monétaire plus forte et plus protectrice ?

: nous ne pouvons nous satisfaire d'une union monétaire qui ne soit pas davantage une union économique. C'est tout l'esprit de la feuille de route dont nous avons discuté avec l'Allemagne. Nous avons prévu de parachever l'union bancaire, de faire en sorte que son filet de sécurité ultime soit pleinement opérationnel, de renforcer encore le mécanisme européen de stabilité et de créer un véritable budget de la zone euro. Il s'agit là de réponses indispensables pour faire émerger une union prospère et plus stable. évidemment, ces propositions doivent être portées au sein de l'Eurogroupe, ce que nous avons commencé à faire. Les autres États membres sont convenus qu'il s'agissait d'une base de travail solide. Il est toutefois normal, et même sain, que des discussions aient lieu. Je puis vous assurer que Bruno Lemaire et Olaf Scholz sont absolument déterminés à convaincre nos partenaires de la zone euro d'avancer. Nous sommes ouverts aux discussions, mais il faut maintenant avancer, et très vite. La parole

Madame la secrétaire d'État, la France est championne- pas encore de football, mais de la dépense publique, au dernier rang des pays de l'OCDE. Le problème n'est pas nouveau : cela fait cinquante ans que les gouvernements successifs se sont essayés à rendre plus efficaces les dépenses de l'État. Si comme moi, vous aimez l'action publique, si vous aimez gagner du temps, vous simplifier la vie et que vous êtes un peu, le sujet va vous passionner. » Ces mots, prononcés par le Premier ministre le 13 octobre 2017, confortaient mon enthousiasme de participer au Comité Action publique 2022. Ce comité, chargé par le Gouvernement de pointer les principaux dysfonctionnements des services publics et de dresser la liste des solutions possibles, devait être celui d'un nouveau monde. Je cite toujours le Premier ministre : « Nous aurions pu faire comme avant présenter un plan d'économies. Nous avons voulu faire quelque chose de radicalement différent, à la fois de plus intelligent, de plus respectueux et de plus durable : transformer en profondeur l'action publique. Au terme des travaux du Comité, mon enthousiasme s'est éteint et l'espoir d'un nouveau monde n'est plus qu'un mirage. Alors que l'implication des membres du Comité a été forte pour essayer de proposer des idées disruptives, pour rendre l'action publique plus efficace par de la simplification, de la rationalisation, de la mutualisation, très rapidement les seules propositions retenues furent celles qui se chiffraient en millions d'euros d'économies. Mes questions sont donc les suivantes, madame la secrétaire d'État. Le rapport du Comité Action publique 2022, et plus largement le programme Action Publique 2022, sera-t-il porté à la connaissance des parlementaires, des élus locaux, voire des citoyens ? Les expériences antérieures ont montré l'inefficacité d'une vision purement technocratique. Quel est le calendrier du chantier Action Publique 2022 ? Quel est le montant réel du plan d'économies ? À quelle échéance ? Les économies porteront-elles sur le budget de l'État ou sur celui des collectivités locales, qui ont déjà largement contribué ?

Nous allons poursuivre

rien dire ! Mon ministère, par exemple, a engagé de façon très détaillée la revue des aides publiques aux entreprises. Il s'agit bien d'une transformation de l'action publique et d'une transformation en profondeur de l'organisation de nos moyens, pour répondre aux missions prioritaires. Ce n'est

La parole est à M. André Gattolin, pour le groupe La République En Marche.

au sommet de l'agenda du Conseil européen qui se tiendra en fin de semaine à Bruxelles. Il y a urgence à définir des règles et des moyens d'action communs. Toutefois, au regard des positions très divergentes en présence, il y a peu de chances qu'un accord unanime soit trouvé. L'Europe doit pourtant impérativement avancer, notamment sur la question de l'accueil des réfugiés, en trouvant une solution au refus des pays de Visegrad d'honorer leurs quotas d'« asilés », fixés à la suite de la crise migratoire de 2015. plusieurs solutions sont évoquées. Très récemment, le Président Macron a suggéré de conditionner l'attribution de certains fonds structurels européens à l'accueil effectif de réfugiés. Si un tel instrument peut se révéler efficace, il nous faudra d'abord inscrire cette conditionnalité de principe dans le prochain cadre financier pluriannuel, ce qui n'est pas encore acquis. Pour autant, ce type de mesure contraignante à l'encontre des États réfractaires devrait utilement s'accompagner de mesures d'ordre plus incitatif. La Commission envisage la création d'une agence européenne pour l'asile, dont les contours demeurent encore peu définis.

peut se retrouver défait en quelques mois ou quelques années. Le Brexit montre que le délitement peut être parfois très rapide. L'Union européenne est soumise en ce moment à des tests de solidité et de souveraineté,

éviter que certains demandeurs d'asile, légitimement éligibles à ce droit, n'aient à faire cette traversée de la mort. C'est tout l'objet des missions

voilà une semaine, douze individus, dont neuf détenus, soupçonnés de trafic international de drogue portant sur des quantités importantes de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, d'ecstasy ou encore de Kétamine, devaient comparaître devant le tribunal correctionnel de Pontoise. Parmi ces individus, prévenus incarcérés ont dû être remis en liberté faute de magistrats disponibles, à la suite de l'arrêt maladie de la juge chargée du dossier, le délai légal de six mois de détention provisoire obligeant à les libérer.

Par ce jeu des actes manqués, notre système s'épuise et se ridiculise. Comment une institution aussi importante que l'autorité judiciaire ne peut-elle être en capacité d'assurer son rôle ? Cette affaire n'a malheureusement rien d'exceptionnel et ne doit pas être banalisée sous prétexte de la crise que subit l'institution. Madame la garde des sceaux, comptez-vous attendre mars 2019- c'est la date qui a été avancée - pour que ces trafiquants passent en jugement ? Plus largement, je souhaiterais savoir comment vous comptez régler au plus vite ces situations, afin qu'elles ne puissent se reproduire. En effet, elles créent un sentiment d'impunité pour les délinquants et de désespérance pour les magistrats, les policiers et les victimes. Prévoyez-vous des mesures explicites afin d'endiguer le phénomène de surcharge de travail Il y va, me semble-t-il, de la crédibilité du système judiciaire et légal français.

Concernant l'affaire qui vient d'être évoquée, j'ai saisi les chefs de cour de la Cour d'appel de Versailles pour leur demander des explications précises sur quatre points. J'ai sollicité des précisions sur l'organisation générale du service correctionnel, notamment sur l'audiencement, que sur l'existence d'un dispositif de remplacement des magistrats en cas d'empêchement. J'ai demandé un rapport circonstancié sur le déroulement de l'audience qui a été évoquée et sur l'impossibilité d'examiner cette affaire avant plus d'un an. J'ai en outre souhaité avoir des éléments d'explication sur les conditions dans lesquelles le renvoi a été prononcé, et s'il a été précédé, comme cela doit être le cas, d'une information à la présidente de la juridiction. J'ai enfin demandé à être éclairée sur les difficultés particulières qui auraient justifié un tel report et une telle situation. En fonction des éléments qui me seront remis, j'envisagerai ou non la saisine de l'Inspection générale de la justice.

mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, les associations jouent un rôle déterminant dans notre pays, notamment au titre de la cohésion sociale. Elles ont été récemment fragilisées par la diminution drastique des contrats aidés, ainsi que par la baisse des subventions qui leur étaient accordées. Aujourd'hui, elles le sont de nouveau, en raison de certaines mesures adoptées dans le cadre du dernier projet de loi de finances. En effet, la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière a fait sortir du calcul de cet impôt nombre de contribuables, qui ont par conséquent perdu la possibilité de bénéficier de la déduction fiscale de 75 % et ont donc interrompu leurs dons.

ailleurs, l'une des principales sources de financement des associations est la multiplicité des petits dons. Or, à la suite de la hausse de la CSG,

À cela vient s'ajouter le fait que la mise en place du prélèvement à la source, qui n'aura pourtant pas de conséquences sur les déductions fiscales, crée une incertitude, voire une confusion, l'année blanche perturbant la campagne de collecte de dons

Certes, le nombre d'assujettis à l'IFI est par nature moins important que le nombre de ceux qui étaient assujettis à l'ISF. C'est le sens même de la réforme. Toutefois, à l'inverse, l'allégement de la fiscalité sur le capital et la redirection de l'épargne pourront être un facteur positif pour les secteurs concernés par les dons. Il faut également rappeler que les anciens donateurs assujettis à l'ISF et qui ne seront pas assujettis à l'IFI sont, dans leur grande majorité, imposables pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Ils pourront donc bénéficier à ce titre de la réduction d'impôt sur le revenu pour dons aux oeuvres, à un taux très avantageux de 66 %.

Je vous remercie

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

heures de débat en séance publique, l'Assemblée nationale vous a passé le relais pour travailler et enrichir un texte clé pour l'agriculture et l'alimentation dans notre pays.

et du sérieux du travail mené par la Haute Assemblée, et plus particulièrement par les rapporteurs. Je note néanmoins que, si vous avez supprimé 18 articles en commission, vous n'avez pas manqué d'en créer 11 nouveaux. Je reconnais là non seulement la sagesse des sénateurs, mais aussi leur grande créativité. Si nous nous retrouvons s'agissant de certaines suppressions d'articles, selon moi justifiées, il n'en demeure pas moins que la disparition de certains articles ou alinéas sera l'objet de discussions, au cours des heures qui nous réuniront autour d'un seul et unique objectif, celui de répondre aux exigences identifiées au cours des États généraux de l'alimentation. Il s'agit de l'urgence à restaurer la capacité des agriculteurs à tirer un revenu décent de leur travail la nécessité de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens en proposant à tous et à chacun une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. Ce projet de loi est le premier outil de la feuille de route de la politique de l'alimentation tracée par le Premier ministre et les ministres présents le 21 décembre dernier, lors de la clôture des États généraux. Mais il n'est pas le seul, et il importe de jouer de la complémentarité de tous les outils pour avancer sur les sujets agricoles et alimentaires Je pense notamment aux plans de filière, qui signent l'engagement des acteurs économiques au programme « Ambition bio 2022 », que j'ai eu le plaisir de présenter hier ; au renforcement de la stratégie relative au bien-être animal ; et à la feuille de route sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante des pesticides, qui témoignent des dynamiques de transformation qui sont à l'oeuvre ; au plan d'action « bioéconomie », qui ouvre des pistes de diversification des revenus agricoles au travail sur la fiscalité agricole, que j'ai engagé avec Bruno Le Maire, des parlementaires et des représentants des acteurs de l'agriculture ; enfin, au volet agricole du grand plan d'investissement, qui marque la volonté de l'État d'être présent aux côtés des acteurs pour accompagner les évolutions en cours ou à venir. La liste, vous le savez, n'est pas exhaustive. Mais il me paraissait important de remettre en perspective le travail que nous conduisons. Nous avons besoin d'un cadre légal clair, facilitateur,

nouvelles. Depuis le début de la semaine dernière, les interprofessions sont une nouvelle fois reçues à mon ministère, afin de faire un point sur la mise en oeuvre des plans de filière, qu'il s'agisse du travail sur la contractualisation- je pense notamment aux indicateurs -ou de l'affinement et de la concrétisation des engagements sociétaux.

Vous le savez, nous devons lutter à la fois contre ceux qui veulent que rien ne bouge et qui se complaisent dans des politiques figées, pour mieux les dénoncer ensuite, et ceux qui veulent absolument imposer leurs visions leurs modèles sans se soucier des difficultés créées. Cette politique du « pied au mur » ne permet pas les démarches de progrès auxquelles je crois et que je souhaite construire avec vous dans un dialogue singulier, permanent et respectueux des valeurs de chacune et chacun. L'agriculture et l'alimentation sont au coeur de notre projet pour la France. Pourquoi ? Parce qu'elles sont l'une des clés de notre souveraineté. Parce que l'agriculture est au carrefour de multiples politiques qui façonnent notre pays l'alimentation, l'aménagement du territoire, la ruralité, la transition écologique, le commerce extérieur et les relations internationales. Parce que l'une des missions premières de l'agriculture est de nourrir la population. Parce que l'alimentation est un enjeu quotidien pour tous nos concitoyens : bien manger, en quantité et en qualité ; permettre à chacun de manger sain, sûr, durable, sans oublier la dimension conviviale de nos repas, qui fait partie des grandes traditions françaises. En abordant cette discussion, nous devons penser tout particulièrement aux agriculteurs et à tous nos concitoyens, comme nous l'avons fait pendant les États généraux de l'alimentation. de l'alimentation. Pensons aux agriculteurs. L'agriculture française doit pouvoir retrouver son esprit de conquête. Les agriculteurs disposent d'un savoir-faire et d'une force de travail indispensables à la vie économique de la France et à l'aménagement de nos territoires. Ils sont les gardiens des paysages et de la biodiversité, au coeur de notre identité et de nos défis alimentaires, économiques et environnementaux. Comment faire réussir la France sans l'agriculture française ? C'est parce que nous voulons une agriculture prospère, compétitive et durable que notre projet vise à soutenir les agriculteurs, afin qu'ils puissent vivre de leur travail, tout simplement. Au travers de ce projet de loi, nous voulons donc défendre avec vous une agriculture riche de la diversité de ses modèles agricoles. Il ne s'agit pas d'opposer ces modèles. Il faut au contraire qu'ils soient complémentaires et créent les ressources suffisantes, pour développer nos économies locales et nous permettre d'être présents sur les marchés nationaux et internationaux. Parce que nous souhaitons, dans notre projet de transformation de la France, que le travail paie, nous devons nous engager pour que les agriculteurs perçoivent le juste prix de leur labeur. Pensons aussi à nos concitoyens. Nous sommes tous sensibles à au moins l'une des facettes du chantier sociétal des États généraux de l'alimentation. Nous sommes attentifs à ce que mangent nos enfants à la maison et à l'extérieur. Nous sommes aussi préoccupés de l'alimentation des personnes les moins favorisées, comme en témoigne la générosité des dons des Français aux associations caritatives. Nous sommes soucieux du bien-être animal. Nous sommes concernés et vigilants sur les enjeux environnementaux. Grâce à ce texte, je veux redonner du pouvoir aux producteurs dans la chaîne de valeur. Nous partageons tous le même constat. La situation n'a que trop duré. Les agriculteurs subissent de plein fouet une guerre des prix et ne dégagent pas, ou plus, les marges de manoeuvre qui sont indispensables, tant à la rémunération de leur travail ou de leur capital qu'à la montée en gamme des productions alimentaires. Cette guerre des prix se nourrit du déséquilibre de l'offre et de la demande, de l'absence d'organisation de la production, de la concentration toujours plus forte du secteur la distribution. Elle se nourrit aussi, parfois, de la défiance des consommateurs et des injonctions contradictoires qu'ils envoient aux producteurs. Je ne crois pas que l'on puisse avoir des productions toujours plus saines, plus élaborées et plus durables avec des prix toujours plus bas et des promotions toujours plus attrayantes. ! Sans nier qu'il y ait eu des parenthèses plus favorables pour certaines productions, le sujet auquel il nous faut apporter des réponses est bien celui de la répartition et de la relance de la création de valeur, pour lutter contre la vente à des prix anormalement bas. Ma priorité est bien de redonner aux agriculteurs le juste prix de leur production et la visibilité indispensable à tout entrepreneur pour penser le temps long et produire ainsi une alimentation de qualité, dans le respect de règles sociales, environnementales et sanitaires renforcées. Que propose aujourd'hui le projet de loi pour atteindre cet objectif ? Le titre I regroupe une palette de dispositifs visant à redonner sa juste place à chaque maillon de la chaîne de valeur agricole et alimentaire la construction du prix à partir de l'amont et des coûts de production des agriculteurs, puisque le contrat et les prix associés seront désormais proposés par celui qui vend la clause de renégociation, plus opérationnelle, pour faciliter la réouverture des négociations commerciales en cas d'évolution des coûts de production ; la lutte contre les prix abusivement bas, des contrôles et des sanctions ; le rôle accru de la médiation ; le renforcement des interprofessions ; le travail sur le statut et le rôle de la coopération agricole ; l'encadrement des promotions ; le seuil de revente à perte, fixé à 10 %. Sur ce dernier point, je souhaite rassurer les consommateurs, parfois inquiets des propos alarmistes de certains distributeurs. Oui, c'est vrai, le relèvement du seuil de revente à perte et la fin des promotions excessives vont induire pour la distribution, dans un premier temps, une hausse de marge et de chiffre d'affaires. Mais non, d'affaires. Mais non, il n'y a aucune fatalité à ce que ces hausses se traduisent par une augmentation globale des prix pour le consommateur ! Chaque distributeur pourra revoir ses marges à la baisse sur d'autres produits, tout en augmentant le prix payé à ses fournisseurs, notamment les producteurs et les PME de l'agroalimentaire. Ce rééquilibrage des marges se répartira sur un nombre si important de produits que le distributeur pourra finalement contribuer à la meilleure rémunération des agriculteurs et préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Vous le voyez, l'édifice du titre I de la loi est un tout, tout, un ensemble cohérent de mesures qui repositionnent chaque acteur sur ses compétences et face à ses responsabilités. À ce sujet, et nous aurons l'occasion d'en rediscuter je ne suis pas en phase avec les dispositions sur l'élaboration des indicateurs dans la version actuelle du projet de loi. Au-delà du risque juridique de la rédaction actuelle, cela revient à fragiliser le rôle des interprofessions et à déresponsabiliser les opérateurs, ce qui est contraire à notre objectif. Nous naviguons, certes, dans un environnement juridique contraint, mais nous ne pouvons pas l'ignorer, au risque de prendre des dispositions qui ne seraient pas opérationnelles et seraient donc sans effet. Il faut que tout le monde en ait conscience. Si chacun, demain, prend ses responsabilités, cette loi sera efficace et opérationnelle. Elle ne laissera pas la place aux interprétations s'agissant de la répartition de la valeur créée. Je suis convaincu- je crois que vous l'êtes aussi sur ces travées -que le premier des défis qui attendent nos modèles agricoles, c'est bien de recréer des marges financières pour offrir à la fois de la visibilité pour investir et transformer durablement nos modèles. Cette visibilité et cette capacité à penser l'agriculture à moyen terme sont indispensables pour conduire les transformations rendues nécessaires par le contexte économique, mais aussi pour répondre aux attentes sociétales. À cet égard, les titres suivants du projet de loi, qui sont à mes yeux aussi importants que le premier, viennent soutenir la première jambe du texte, à savoir la finalité de la production agricole, l'alimentation des Françaises et des Français. Bien plus qu'un besoin élémentaire- les États généraux l'ont souligné -, la consommation de denrées alimentaires est un acte auquel nos concitoyens accordent un sens profond, une attention renforcée, presque politique, au sens noble du terme.

Le projet de loi traduit la volonté du Gouvernement de porter une politique alimentaire favorisant des choix qui préservent le capital de santé de chacun et le capital environnemental de tous. En matière de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, le projet de loi interdit les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits. Je souhaite que nous puissions rouvrir ce débat

les pouvoirs d'enquête et de contrôle des agents chargés de la protection de la santé, de la protection animale et de la sécurité sanitaire des aliments sont renforcés. Pourquoi ? Pour accroître l'efficience des contrôles de l'État. Dans le domaine du bien-être animal, le texte initial du Gouvernement prévoyait déjà d'étendre le délit de maltraitance animale, ainsi que le doublement des peines en cas de délit constaté lors de contrôles officiels. proposé de donner la possibilité aux associations de protection des animaux de se porter partie civile en cas d'infraction constatée par un contrôle officiel. Je me félicite que cet article ait été voté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Autre volet clé du projet de loi, à l'intérieur du titre II, le Gouvernement veut faire de la politique de l'alimentation un moteur de réduction des inégalités sociales. Nous le savons tous, l'accès à une alimentation variée et de qualité est encore aujourd'hui très corrélé à l'appartenance à une catégorie sociale. C'est le cas de Pour tenter de réduire ces inégalités sociales, il vous est proposé, à l'article 11, de faire de la restauration collective un levier d'amélioration de la qualité de l'alimentation pour tous, et ce dès le plus jeune âge. Comment ? La restauration collective publique représente plus de la moitié des 7,3 milliards de repas hors foyers servis en France chaque année. Nous souhaitons que la restauration collective publique s'approvisionne avec au moins 50 % de produits issus de l'agriculture biologique, locaux ou sous signes de qualité à compter du 1 janvier 2022. Sur ce point, je me félicite que vos rapporteurs aient proposé de réintroduire l'objectif d'atteindre 20 % de produits issus de l'agriculture biologique d'ici à 2022. Enfin, le projet de loi vise à lutter contre la précarité alimentaire et à limiter les conséquences environnementales du gaspillage. Les articles 12 et 15 ont donc pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective par la mise en place d'un diagnostic obligatoire et d'étendre à la restauration collective et à l'industrie agroalimentaire le don alimentaire.

Je serai bien entendu attentif à vos propositions pour améliorer le texte. Il s'agit de nous inscrire collectivement et résolument dans une trajectoire qui respectera tant les hommes, du producteur au consommateur, que l'environnement dans lequel ils évoluent. Construire une trajectoire pour tirer notre agriculture vers le haut, par l'innovation, par l'investissement, par la montée en gamme, par la confiance, c'est lui donner toutes les chances de résister aux défis de la mondialisation. Avec le Président de la République et le Premier ministre, je veux refonder le pacte social entre les agriculteurs et la société pour leur redonner la fierté de leur travail et redonner à la France la fierté de son agriculture. La parole est à M. le rapporteur.

pour le Sénat d'examiner le projet de loi qui en résulte. Ce texte prétend créer les conditions d'augmentation des revenus des producteurs. C'est une légitime priorité nationale. Comment peut-on en effet assurer

et bénéficier de la même modernité que dans les autres pays européens. Monsieur le ministre, soyez assuré que vous trouverez toujours un soutien appuyé dans la Haute Assemblée dès qu'il s'agira d'assurer une meilleure rémunération de nos agriculteurs, actifs ou retraités. De nombreuses filières souffrent d'une guerre des prix toujours plus vivace. Les revenus des producteurs n'ont pas à financer les promotions des consommateurs. Tout ce qui permettra aux producteurs de mieux peser dans la chaîne de valeur d'un produit est essentiel. Tout ce qui permettra aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier recevra notre aval. Toutefois, ce projet de loi prend un risque immense : celui de ne rien changer pour nos agriculteurs. Car, après tant de promesses semées par le Président de la République et par le Gouvernement,

on peut considérer que seulement 40 % des producteurs seront concernés par le texte. Deuxièmement, le projet de loi ne parle que du prix, qui n'est qu'une composante du revenu. Il ne parle ni des charges, ni de la fiscalité, ni des aléas climatiques et économiques, ni des autres sources de revenus, comme la politique agricole commune. À cet égard, monsieur

nous semble-t-il, en train de perdre les négociations sur le budget de la politique agricole commune à Bruxelles ! Ces négociations se traduiront directement, et de manière certaine, par une baisse des revenus aux producteurs, puisque c'est une partie de leur chiffre d'affaires.

Il est même possible que le projet de loi fasse l'inverse de ce qu'il prétend. C'est un pari, monsieur le ministre. Et ce pari très risqué pourrait se retourner contre les producteurs. Je suis

La commission a considérablement renforcé les armes des producteurs dans leurs négociations, en instaurant une procédure de saisine au fond du juge en cas d'échec de médiation. Nous avons aussi instauré certains produits spécifiques. Nous avons prévu une pleine application du droit français des pratiques anticoncurrentielles aux négociations effectuées à l'étranger. Nous avons imposé de formaliser par écrit et de motiver le refus de certaines conditions générales de vente par un distributeur.

Cela implique qu'eux-mêmes et leurs familles puissent vivre décemment de leur travail et qu'ils soient accompagnés dans la recherche de débouchés rémunérateurs et la montée en gamme de leurs productions, afin de répondre aux attentes nouvelles des consommateurs. Les liens de causalité entre la première et la seconde partie du texte sont donc évidents. Ils se sont parfois trouvés malmenés, au fil des débats à l'Assemblée nationale, à mesure que des sujets divers et induisant de nouvelles charges pour l'agriculteur étaient introduits. Monsieur le n'y a-t-il pas une certaine forme de schizophrénie à chercher, dans une première partie, à augmenter les recettes des agriculteurs et à créer, dans une seconde, des contraintes nouvelles, aboutissant à reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre ? C'est cet écueil que notre commission a tenté d'éviter, en se concentrant sur l'objectif essentiel de ce projet de loi, dans un contexte- il faut le souligner -de grand désespoir et d'impasse pour de nombreux agriculteurs français, qui en attendent beaucoup. l'exercice est délicat, car il amène à reporter certains débats sur des sujets, comme le bien-être animal, éminemment préoccupants et importants, mais qui ne sont pas à leur place dans un projet de loi, dont, encore une fois, l'objet essentiel est la survie de notre agriculture de notre agriculture et la prédominance du modèle des exploitations françaises. C'est en ce sens, et par cohérence avec les espoirs nés des États généraux de l'alimentation, que nous avons cherché à recentrer le texte. Monsieur le ministre, je regrette que le Gouvernement revienne sur bon nombre des propositions avancées par notre commission, en rétablissant presque systématiquement la rédaction de l'Assemblée nationale. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a, semble-t-il, déjà fermé la porte à tout accord en commission mixte paritaire. Mais nous espérons que la voie de la sagesse et du dialogue parlementaire reprendra le dessus. En matière d'alimentation, la commission a cherché à adapter la loi aux réalités du terrain, notamment s'agissant des obligations nouvelles faites à la restauration collective publique concernant l'approvisionnement local et de qualité. En ce sens, je vous proposerai des assouplissements pour les gestionnaires, une plus grande structuration des approvisionnements locaux permettant de répondre à l'objectif des 20 % de produits bio, auquel nos filières locales et nationales ont confirmé pouvoir répondre. La commission a effectivement ajouté quelques dispositions, mais c'est pour mieux protéger et promouvoir les productions françaises, qu'il s'agisse du vin, avec une obligation d'information sur l'origine dans tous les établissements qui en vendent et le maintien d'une déclaration de récolte obligatoire, ou encore du miel. Elle a aussi « toiletté » le texte d'un certain nombre de dispositions « bavardes » ou redondantes, qui n'apportaient rien au droit existant. En matière de bien-être animal, la commission a jugé que l'équilibre auquel sont parvenus nos collègues députés, consistant à responsabiliser les filières et leur faire prendre des engagements, ne devait pas être remis en cause. Le champ des infractions de maltraitance animale pour lesquelles des associations pourraient se porter partie civile a donc été bien circonscrit. De même, les modalités retenues pour expérimenter la vidéosurveillance dans les abattoirs volontaires ou tester les abattoirs mobiles constituent des avancées. Sur la partie relative aux produits phytopharmaceutiques, la commission n'a pas voté les mesures sur lesquelles elle manquait d'informations. L'étude d'impact relative à l'interdiction des remises, rabais et ristournes figurant à l'article 14 se résume à une page de considérations peu étayées ou chiffrées. De même, la demande d'habilitation à légiférer pour séparer les activités de vente et de conseil est très vague, vague, le projet du Gouvernement n'étant pas défini. La commission a évité tout surcroît de charges qui ne se justifierait pas. Elle est ainsi revenue sur l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur la vente de produits phytopharmaceutiques, sachant que, en la matière, c'est non pas le prix qui fait l'usage, mais bien la nécessité de traitement. Elle a souhaité l'émergence d'un conseil individuel véritablement stratégique et pluriannuel, permettant d'accompagner l'exploitant, pour lui permettre d'optimiser à moyen terme ses usages de produits phytopharmaceutiques. Pour ce conseil, l'incompatibilité avec les activités de vente de produits phytopharmaceutiques En matière de réduction des usages des produits phytopharmaceutiques, toutes les initiatives favorisant l'émergence de solutions de remplacement sont valorisées. Seront mises en place des procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle, la procédure d'évaluation de la toxicité du produit étant maintenue, conformément à la réglementation européenne. Les préparations naturelles peu préoccupantes, ne figurant pas déjà dans la liste préétablie, bénéficieront d'une évaluation simplifiée. Les progrès technologiques, comme l'agriculture de précision, constituent de formidables leviers pour nos agriculteurs. En ce sens, la commission a élargi le champ de l'expérimentation de l'épandage par drones, sur les terrains les plus dangereux, présentant une pente supérieure à 30 %, y compris pour les produits phytopharmaceutiques. Enfin, en matière d'énergie, la commission a marqué son soutien aux démarches de diversification et de production d'énergies renouvelables par les agriculteurs, en consolidant le droit à l'injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturel situés à proximité d'un méthaniseur, y compris lorsqu'il n'est pas dans le périmètre d'une concession, afin que la mesure ait réellement un sens. Pour conclure, la commission a donné un contenu au volet simplification des normes agricoles, en consacrant l'existence juridique du comité de rénovations des normes en agriculture, qui produira prochainement un rapport sur la surtransposition en agriculture. En bref, la commission des affaires économiques du Sénat accompagne la montée en gamme des productions, favorise de nouveaux débouchés pour les produits locaux de qualité, tout en assurant une meilleure maitrise des produits phytopharmaceutiques et une attention aux conditions de bien-être animal, sans pour autant déséquilibrer encore une agriculture française en recherche de compétitivité dans un environnement de plus en plus concurrentiel. La parole

Au-delà des affrontements stériles et dépassés entre les enjeux économiques, sanitaires et environnementaux, nous devons trouver des solutions équilibrées et pérennes sur ces sujets.

De même, nous ne pouvons pas méconnaître les difficultés des agriculteurs, qui aspirent à vivre correctement de leur métier, et avec dignité. Guidée par ce souci d'équilibre, notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie de trente-neuf articles du présent projet de loi, sur trois thèmes : la restauration collective, le gaspillage alimentaire et les produits phytopharmaceutiques. Outre vingt-huit articles examinés pour avis, onze ont fait l'objet d'une délégation au fond de la part de la commission des affaires économiques. Nous avons appréhendé ces sujets avec pragmatisme, en privilégiant l'accompagnement des acteurs et la définition d'objectifs atteignables à des échéances raisonnables, plutôt que de proposer des ruptures brutales. Face aux nombreuses mesures adoptées par l'Assemblée nationale, nous avons également veillé à la qualité du projet de loi, en distinguant les dispositions qui contenaient de réelles avancées de celles qui relevaient davantage d'un signal purement politique. Permettez-moi à ce titre de déplorer fortement, monsieur le ministre, que le Gouvernement ait déposé de très nombreux amendements de suppression des modifications introduites en commission sur l'ensemble du projet de loi. Il y a là un signal inquiétant sur l'attention que vous accordez au travail parlementaire et au bicamérisme. Très bien ! J'en viens aux modifications apportées au texte sur l'initiative de notre commission. Je souhaiterais, tout d'abord, exprimer ici mes inquiétudes concernant l'article 11, qui fixait initialement deux objectifs ambitieux sur les produits servis en restauration collective, en visant 50 % de produits « sous signe de qualité », dont 20 % de produits issus de l'agriculture biologique. Cet objectif de 20 % a été supprimé par la commission des affaires économiques, ce qui envoie un signal négatif par rapport aux fortes attentes de la population dans ce domaine. Nous devons absolument soutenir la présence de produits bios issus des exploitations disposant de la certification « haute valeur environnementale » ou du commerce équitable, en privilégiant bien sûr les productions françaises. Les Chinois, concurrents redoutables au niveau économique, ont bien perçu l'ouverture de ce nouveau marché et sont déjà prêts à répondre à cette demande grandissante. Il convient Il faudra plus que des paroles et des actes, monsieur le ministre : il faudra des engagements forts du Gouvernement pour soutenir la conversion de nombreuses exploitations si l'on veut parvenir à l'objectif de 15 % de la surface cultivée en bio. l'aménagement du territoire et du développement durable a souhaité prévoir une évaluation scientifique des risques sanitaires liés à l'utilisation des contenants alimentaires dans les cantines ; nous avons introduit une interdiction des pailles. S'agissant de l'interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines, de nombreux amendements de suppression ont été déposés. Nous aurons bien sûr un débat sur ce point.

Sur le gaspillage alimentaire, notre commission a souhaité maintenir la mise à disposition des aux seuls clients qui en feraient la demande pour emporter chez eux les restes de leur repas. Nous avons, en outre, prévu l'utilisation de contenants réutilisables ou recyclables dans le cadre de la vente à emporter. Enfin, notre commission a envoyé des signaux clairs pour réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides, sans pour autant priver brutalement leurs utilisateurs de solutions face aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.

Premièrement, sur l'insertion en commission d'une dérogation inappropriée au dispositif « zéro phyto » dans les espaces verts des collectivités territoriales. Deuxièmement, sur la suppression de la disposition permettant de conforter l'interdiction d'utiliser des produits contenant des néonicotinoïdes, adoptée dans la loi biodiversité. Nous avions proposé en commission de renforcer de rôle de l'ANSES, seule habilitée à prendre des décisions crédibles. sur la nécessité de permettre au préfet, lorsque les circonstances locales le justifient, d'encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de zones habitées. Je conclurai en rappelant que l'avenir de notre agriculture et de notre alimentation est l'affaire de tous, et que la transition vers un modèle agricole plus durable ne pourra s'effectuer que par le biais d'un partenariat constructif. J'espère que nos débats contribueront à apporter des réponses crédibles, mais ambitieuses, à ces défis. La parole

Cette exigence revêt plusieurs sens. Bon gré, mal gré, il nous faut, à travers les divergences et les désaccords, bâtir un nouveau modèle agricole qui soit économiquement viable et écologiquement responsable. Ces prochains jours, l'hémicycle sera le terreau de discussions passionnantes soulevées par l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Permettez-moi de saluer tout particulièrement le travail remarquable

Edgard Pisani le disait déjà dans les années soixante, l'agriculture est l'expression de l'état d'une société. Parce qu'elle concerne chacun d'entre nous, elle est la traduction des questions fondamentales touchant au rapport de l'homme à la terre et au vivant. L'agriculture est plus que la partie d'un ensemble. C'est une question sociale, environnementale, de santé, de ruralité ou encore technique. Pour toutes ces raisons, l'agriculture est un sujet éminemment politique, catalyseur de toutes les divergences. Le débat soulève un certain nombre de contradictions apparentes, qu'il va nous falloir dépasser, entre quantité et qualité, circuits de proximité et mondialisation, progrès économique et responsabilité sociétale, tradition et modernité, pour n'en citer que quelques-unes. Je suis certain que nous saurons faire preuve d'inventivité, de discernement et de bienveillance tout au long du débat, pour permettre à la politique agricole de s'adapter aux évolutions de la société, tout en préservant les plus fragiles des dommages économiques que pourraient causer ces évolutions. Le progrès environnemental est au coeur des préoccupations de la société et le groupe Les Indépendants - République et Territoires partage cette sensibilité. Cependant, il nous faut veiller à aménager des marges de manoeuvre suffisantes pour les agriculteurs dont les revenus sont les plus précaires. Pour certains, la situation est telle que les marges nettes dégagées ne leur permettent pas de couvrir les coûts de production. Les distributeurs se livrent à une guerre des prix depuis 2013, ce qui fragilise l'ensemble de la filière. Pour répondre à cette problématique, le texte vise à renverser la logique de construction des prix pour permettre une meilleure prise en compte des coûts de production et une plus juste rémunération des producteurs en plaçant ceux-ci au centre des négociations, et en fixant un ensemble d'indicateurs pertinents. Nous espérons que ces dispositions mettront fin à la guerre des prix livrée par ces gens qui, pour reprendre les paroles d'Oscar Wilde, « savent le prix de tout et ne connaissent la valeur de rien Nous vivons en France, avec l'assurance de manger à notre faim, pas seulement aujourd'hui ou demain, mais pour le restant de nos jours. C'est vrai pour la plus grande majorité des Français. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, le texte prévoit de nouveaux leviers, afin de lutter contre la précarité alimentaire et développer la pratique du don. Autre versant du texte, la lutte contre le gaspillage alimentaire est un sujet qui mérite toute notre attention. J'avais déjà déposé une proposition de loi contre le gaspillage alimentaire en 2015 à l'Assemblée nationale. Je vous proposerai une nouvelle disposition visant à fixer un objectif non contraignant de réduction des restes alimentaires. La question alimentaire en France n'est plus uniquement celle de la quantité ; elle est aussi celle de la qualité. Le sociologue Claude Fischler décrit un phénomène de « boîte noire » concernant l'alimentation. On ne sait plus ce que l'on mange ni pourquoi on le mange. Aussi les scandales sanitaires, tels que la fraude à la viande de cheval en 2013, font-ils figure d'électrochocs. Sans tomber dans une information anxiogène, il revient aux pouvoirs publics de permettre au citoyen de décider en âme et conscience de ce qu'il mange. La transparence en matière d'étiquetage est devenue incontournable.

Ces dispositions sont les prémices d'une longue bataille à mener contre le bas de gamme en matière d'alimentation. Pour ouvrir cette boîte noire, nous proposons de rétablir le lien entre le consommateur et le producteur. Je défendrai un amendement d'appel tendant à favoriser le développement des circuits de proximité dans la restauration collective. Cette disposition est aujourd'hui incompatible avec le droit européen, mais celui-ci n'est pas immuable : il peut encore évoluer, sous l'influence des aspirations locales. Il revient à la politique de prévoir l'avenir. Or il n'y a nul avenir de l'homme sans respect de la terre et de la biodiversité. Michel Serres disait : « J'enchante ce paysage qui me fait. Agriculture et paysage sont deux versants d'une même réalité. Nous proposerons deux amendements visant à limiter l'artificialisation des sols et incitant l'État à prendre ses responsabilités en matière de déforestation importée. En matière de bien-être animal, permettez-moi de vous rappeler deux évidences : l'animal est non pas une chose, mais un être vivant ; les agriculteurs ne sont pas des assassins. Aussi nous faut-il veiller à ce que l'homme n'inflige pas aux animaux des souffrances inutiles, sans pour autant stigmatiser le personnel des abattoirs. Tout à fait ! En 1970, un agriculteur couvrait les besoins alimentaires de trois ou quatre personnes. En 2010, il en nourrit une centaine. Évitons au monde agricole de faire le grand écart entre petites fermes et grandes firmes, entre permaculture et monoculture. Il reste tout un monde agricole intermédiaire à réinventer. agronomique, l'INRA, développe en ce moment des expériences sur les associations de cultures pour favoriser la résistance des plantes aux maladies. Nous avons besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. Nous aurons également besoin de faire preuve d'une grande ingéniosité pour maîtriser les réserves d'eau potable, car l'agriculture est consommatrice des deux tiers de cette précieuse ressource. C'est pourquoi la mise en oeuvre d'une stratégie de gestion active de l'eau dans l'agriculture est une priorité. L'agriculture est une science vieille de 10 000 ans, et elle n'a pas fini d'évoluer. Si nous devons libérer l'innovation, moteur de changement, il nous faut aussi prévoir des transitions pour que la révolution agricole à venir soit la plus acceptable possible. La parole est à M. Franck Menonville.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, faut-il rappeler ici le poids économique et stratégique de notre agriculture ? Pourvoyeuse de milliers d'emplois directs et induits, garante d'une alimentation de qualité et de notre indépendance alimentaire, l'agriculture concentre des enjeux fondamentaux, mais elle est aussi un secteur fragile, soumis à différents aléas.

Les États généraux de l'alimentation, organisés sur l'initiative du Président de la République, ont rassemblé autour de la même table tous les acteurs du monde agricole, de l'amont à l'aval. Fruit de ces discussions, le projet de loi soumis à notre examen à partir de ce soir suscite beaucoup d'attentes. La profession agricole observe en particulier avec intérêt le volet sur l'équilibre des relations commerciales. On la comprend Peut-on encore tolérer que les agriculteurs soient la variable d'ajustement de la guerre des prix, alors que l'on assiste depuis trop longtemps à une captation de la valeur à leur détriment ? On ne peut, d'un côté, demander aux agriculteurs de répondre aux nouvelles exigences sociétales,

la construction du prix autour d'indicateurs ou encore du relèvement du seuil de revente à perte, le titre I du projet de loi ambitionne un rééquilibrage des relations commerciales,

Il faudra aussi traiter le problème de la concentration des centrales d'achat, en intégrant toutefois leurs propres défis, notamment l'émergence des géants du numérique. Il faut également s'attaquer à l'organisation insuffisante des exploitants autour de structures communes de producteurs et de commercialisation, qui est l'une des conditions importantes d'une négociation commerciale plus équilibrée, le droit européen le permettant. Le projet de loi s'attache aussi à répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité des produits. Il y aura un équilibre à trouver au sein du titre II sur certaines mesures, pour compenser l'excès de zèle des députés et quelques suppressions survenues en commission. Bien sûr, nous souscrivons à une restauration collective de qualité garantissant l'approvisionnement local. Nous sommes également favorables à une réduction progressive des produits phytosanitaires, à condition que des solutions de et que du temps soit donné aux exploitants pour qu'ils puissent s'adapter en s'appuyant sur des arguments scientifiques. À cet égard, le rôle de l'ANSES est fondamental. Le RDSE est sensible au bien-être animal, tant que l'on ne tombe pas dans une radicalité qui aboutirait à créer des normes insupportables pour nos agriculteurs. Très bien ! C'est très vrai ! Évitons donc toute surtransposition de normes européennes. Mes chers collègues, nous avons rendez-vous avec l'avenir de notre agriculture et de nos agriculteurs, qui placent beaucoup d'espoirs dans ce texte, même si nous savons qu'il n'est qu'une facette de la politique publique agricole. Néanmoins, les questions plus générales de la compétitivité et de la réforme fiscale restent en suspens et en réflexion. En attendant, le Sénat doit se mobiliser pour garantir des perspectives à nos agriculteurs, qui sont essentiels au maintien des exploitations et à la vitalité de nos territoires ruraux. La parole est

Ce projet de loi que nous examinons porte une réforme ambitieuse pour l'agriculture française, une agriculture qui permette aux producteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes,

Cette transformation est nécessaire, car le modèle dans lequel nous nous sommes aujourd'hui enfermés n'est pas soutenable : le solde extérieur de l'agriculture reste certes positif, mais il est passé de 12 milliards d'euros à 8 milliards d'euros. Les Français doutent de leur alimentation, nous devons aujourd'hui leur apporter des réponses positives. Nous devons repenser une nouvelle France agricole si nous ne voulons pas que les agriculteurs disparaissent et si nous souhaitons leur permettre de viser des marchés d'excellence, en France et à l'export. C'est le coeur de ce projet de loi, et c'est l'objectif de son titre I. Pour réussir cette montée en gamme, deux conditions s'imposent à nous et surtout aux acteurs du secteur, qui doivent être accompagnés : inverser le rapport de force dans les négociations commerciales ; inciter les interprofessions à prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'elles ont d'ailleurs commencé à faire en présentant chacune son plan de filière. Enfin, les nouvelles attentes des consommateurs sont au coeur du renouvellement de notre modèle agricole et alimentaire. le titre II du projet de loi ouvre la voie à la construction d'une véritable éthique de l'alimentation, assortie d'un pacte pour la préservation de l'environnement et pour le respect du bien-être animal.

la commission remet totalement en cause l'esprit même du texte, qui est de responsabiliser les acteurs et de renforcer le rôle des interprofessions. Elles sont un lieu de concertation. Leur fonctionnement par consensus garantit leur légitimité dans l'exercice des missions que nous souhaitons leur confier.

Si nous ne persévérons pas dans les engagements que vous avez pris, monsieur le ministre, et dans le travail entamé par nos collègues députés, on ne retiendra de ce projet de loi que des débats enflammés, qui auront nourri les colonnes des quotidiens sans faire avancer les choses, comme cela a été le cas à l'issue du débat à l'Assemblée nationale. Non, mes chers collègues, la première mission de ce projet de loi est bien d'équilibrer les relations commerciales et de rendre un revenu digne à nos agriculteurs. Ce texte doit nous permettre de revenir à ce pacte de confiance fondé sur une responsabilité partagée de la fourche à la fourchette, dans la droite ligne des États généraux de l'alimentation et des engagements pris par le chef de l'État. L'esprit de la loi ne fera pas tout, nous en avons conscience ; il faudra que celle-ci soit accompagnée d'autres mesures pour atteindre nos objectifs. Vous avez cité, monsieur le ministre, le Plan « ambition bio », publié il y a quelques jours, et la feuille de route 2018-2022 pour une politique de l'alimentation, en concertation avec les filières. Mais la réforme doit offrir au monde agricole des opportunités de court, moyen et long termes, afin qu'il puisse s'organiser et prendre en main son destin collectivement et en bonne intelligence. Cette réforme doit permettre à chaque citoyen de devenir un consommateur responsable et éclairé.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, longtemps évoqués comme un phénomène principalement urbain, la précarité, la pauvreté et l'exclusion n'épargnent ni le milieu rural ni la population agricole, car il y a aujourd'hui 26,4 % de ménages pauvres chez les agriculteurs et les salariés agricoles. Ces chiffres, nous nous les répétons depuis trop longtemps. Pourtant, rien ne change Nous connaissons les causes principales de cette paupérisation de la majorité des agriculteurs et salariés agricoles de notre pays. Les réformes successives au niveau européen de la PAC et de ses déclinaisons nationales, notamment sous la pression des accords de l'OMC, ont fait de la concurrence libre et non faussée un objectif prioritaire de l'organisation des échanges et ont conduit à la disparition des mécanismes de régulation des prix et des productions. l'échelon national, les agriculteurs, mais aussi les consommateurs, sont devenus une simple variable d'ajustement dans la guerre des prix à laquelle se livrent la grande distribution et les groupes industriels agroalimentaires. Guerre qui déséquilibre la chaîne de valeurs, sape la cohésion sociale et fragilise l'ensemble du secteur agroalimentaire français, pourtant stratégique pour l'économie nationale en termes d'emplois, de balance commerciale, mais aussi de structuration de notre territoire. loi de modernisation de l'économie, nous nous opposions à la libéralisation des relations commerciales au vu de la structuration de la filière agroalimentaire, avec une concentration excessive des centrales d'achat, un tissu de PME éparpillé et des producteurs peu organisés. À l'époque, nous dénoncions une contractualisation qui ne pouvait être gagnante pour toutes les parties, car elle était laissée au seul jeu des forces du marché. N'en déplaise à certains, sans un minimum d'équité contractuelle, aucun marché ne peut fonctionner. Nous n'avons eu de cesse de proposer la mise en place d'outils permettant une meilleure structuration des filières, afin d'assurer une plus grande transparence dans la formation des prix au stade de la production, de la transformation et du commerce. Pour cela, nous proposions une identification claire des marges de chacun des acteurs et une meilleure information des consommateurs, pour les aider à concilier leurs contraintes budgétaires et la qualité de leur alimentation. Nos propositions n'ont pas été acceptées. Depuis lors, le législateur n'a cessé d'intervenir pour tenter de restaurer « la loyauté » ou « l'équilibre » des relations commerciales, sans jamais parvenir à transformer les rapports de force. Les grands distributeurs ont en effet toujours su s'adapter aux nouvelles contraintes. Le texte dont nous débattons aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Comme cela a été rappelé, ce projet de loi est très en deçà des attentes des agriculteurs, loin de la problématique d'un renforcement réel du revenu paysan. Puisque nous discutons des agriculteurs et de l'intervention de l'État, vous me permettrez d'avoir un mot pour les retraités agricoles, qui ne voient toujours pas venir l'augmentation de leur pension de retraite, alors qu'ils vivent bien en dessous du seuil de pauvreté. Nous attendons toujours un signe.

Il est étonnant de voir autant de girouettes, alors que l'hémicycle est assez isolé des courants d'air qui traversent le palais du Luxembourg ! Il faut dire cela à d'autres ! Certes, les contrats seront désormais proposés par les producteurs ou par leurs organisations, plutôt que, comme auparavant, par les acheteurs, mais il est très difficile de mesurer l'impact de cette disposition. Certes, il y a la reconnaissance de la nécessité d'indicateurs plus fiables, mais il y a aussi, dans le même temps, le refus que les indicateurs de coûts de production soient publics. Certes, il y a un renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales, mais, dans le même temps, la possibilité de médiation privée reste ouverte. Certes, il y a un renforcement de l'office d'évaluation des prix et des marges et des interprofessions, mais toutes ces mesures laissent le sentiment d'un travail inachevé. Certes, il y a un relèvement de 10 % du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires, est fondé sur « le seul espoir que cela ruisselle jusqu'aux producteurs ». Et si l'espoir fait vivre, il ne modifie en rien les rapports de force. La majorité des organisations agricoles que nous avons auditionnées ne s'y trompent pas : ce texte ne changera les choses seulement à la marge, car il reste inscrit dans un modèle économique qui favorise le plus fort. Voilà pourquoi nous continuerons à porter la nécessité de prix planchers. Voilà pourquoi nous demandons l'intervention publique, sous la forme du déclenchement d'un encadrement des marges de la distribution en cas de crise. Voilà pourquoi nous proposerons l'interdiction de la revente à perte, la définition d'un prix abusivement bas et la prise en compte du revenu paysan dans la construction des indicateurs Dans son volet « alimentation », le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale était porteur de promesses, mais il aurait été opportun de dédier à cette seconde partie un véhicule législatif propre. Sans surprise, nous regrettons que la commission des affaires économiques du Sénat soit revenue sur des mesures phares. Je n'en ferai pas ici une liste exhaustive, nous y reviendrons dans le cours débat. Ces mesures, loin d'être des contraintes, sont aujourd'hui nécessaires, car elles répondent à une demande sociétale très forte, mais aussi à la nécessité de rétablir la confiance entre les agriculteurs et les consommateurs. Elles répondent également à la nécessité de réorienter notre modèle de production, mais elles répondent surtout à des enjeux de santé publique pour les agriculteurs, les salariés agricoles et les consommateurs. En résumé la philosophie de ce texte, tant dans sa version initiale qu'après passage en commission au Sénat, est ne rien imposer, continuer à faire confiance aux grandes entreprises agroalimentaires et remettre entre les mains des filières la responsabilité de la transition environnementale. Nous sommes loin, très loin, des débats et des conclusions des États généraux de l'alimentation,

encore une fois, de la trahison de cette consultation, qui se disait ouverte et participative. Cette loi n'apportera aucune solution concrète. En l'état, notre groupe ne votera pas ce texte. La parole est

permettez-moi de saluer la méthode et l'organisation des États généraux de l'alimentation, qui ont eu le mérite de mettre tous les acteurs du monde agricole, des producteurs jusqu'à la distribution, autour d'une même table, afin de dresser un constat. Ils ont peut-être aussi permis à chacun de comprendre l'autre pour préserver ensemble une agriculture française de qualité. lors de la présentation de ce projet de loi en conseil des ministres, vous avez développé trois axes : assurer la souveraineté alimentaire ; promouvoir des choix alimentaires au service de la santé ; réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité et durable. Assurer la souveraineté alimentaire, c'est être certain que demain il y aura suffisamment d'agriculteurs qui pourront vivre de leur métier. Promouvoir des choix alimentaires en termes de santé, c'est avoir une volonté de changer de paradigme, c'est prévenir au lieu de guérir. Réduire les inégalités d'accès à une alimentation saine et durable, c'est poursuivre le chemin tracé par Stéphane Le Foll, entamé dans la loi d'avenir vers l'agroécologie, qui doit devenir un modèle agricole. Le titre I du texte a pour ambition de redonner de la valeur au travail des agriculteurs, de donner aux organisations professionnelles les moyens d'exercer toutes leurs responsabilités pour la prise en compte des indicateurs des coûts de production et la construction du prix de vente. C'est une excellente chose, mais les coûts de production peuvent varier pour la même filière d'une région à l'autre. C'est pourquoi nous vous proposerons de prendre l'Observatoire de la formation des prix et des marges comme garant. Les organisations professionnelles doivent être suffisamment représentatives pour assurer les lourdes tâches qui leur seront attribuées dans la négociation avec les transformateurs et les distributeurs, qui, eux, ne manquent pas d'expertise dans ce domaine. Nous vous proposerons d'élargir l'expérimentation des contrats tripartites pour que chacun puisse être payé dignement, mais surtout en toute transparence. L'encadrement des promotions est une bonne chose, comme le relèvement du seuil de vente à perte, fixé à 10 %. Monsieur le ministre, nous savons tous la responsabilité des acteurs de la grande distribution dans la stratégie de guerre des prix incessante à laquelle ils se livrent depuis longtemps et qui a mis à genoux une grande partie de notre agriculture. Permettez-moi de douter que se produise la fin de cette guerre. Je crains que la grande distribution n'hésite pas à importer de la marchandise à moindre coût et à poursuivre ses pratiques. Nous le disons : ce que nous souhaitons avant tout, c'est le juste prix pour tous, de l'agriculteur au consommateur. Mesurant la toute-puissance de la grande distribution, je demeure très dubitatif sur le fait qu'elle veuille aller dans votre sens. Sur les articles suivants, nous sommes d'accord avec vous concernant la restauration collective et l'approvisionnement à hauteur d'au moins 50 % de produits issus de l'agriculture de produits locaux ou sous signe de qualité. Nous nous félicitons également de la réintroduction dans le texte de l'exigence de 20 % de bio. Je sais que la majorité sénatoriale avait fait valoir son désaccord lors de l'examen de la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation. Heureusement, elle évolue, très timidement. Mes chers collègues, vous le savez très bien, c'est une volonté sociétale à laquelle vous ne pourrez pas vous soustraire, et je me félicite d'entendre quelques responsables de la Fédération nationale des syndicats Il est prévu de séparer la vente du conseil pour ne pas être juge et partie. Même si nous avons quelques craintes quant aux coûts supplémentaires engendrés pour l'agriculteur, nous y sommes favorables. En revanche, sur l'interdiction des rabais et des ristournes, certes nous parlons de produits dangereux, monsieur le ministre, je suis certain que cela n'a absolument rien à voir avec la diminution de la consommation. Ces produits sont homologués pour des doses à l'hectare. Ce n'est pas parce que l'agriculteur, en morte saison, va acheter un produit moins cher qu'il va en répandre davantage par la suite.

Bien d'autres sujets seront traités pendant ce passionnant débat. Mais, vous le comprenez, au-delà des lois votées par le Parlement français, un sujet délicat est celui de la réciprocité des normes de production et de qualité. Nous la voulons de la part de tous les pays dont nous importons des produits agricoles, ainsi que de tous les pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange, comme cela a été signifié d'ailleurs dans une récente proposition de résolution sénatoriale sur la Oui, j'en suis convaincu, nous devons produire une alimentation de qualité, saine et durable. Nos agriculteurs n'ont pas peur de la concurrence, car ils savent que la tradition française est empreinte d'un savoir-faire reconnu. En revanche, et j'y insiste, ils veulent se battre avec les mêmes règles. Monsieur le ministre, quand nous imposons à nos agriculteurs de nouvelles normes, tous les produits importés doivent s'y conformer ; c'est nécessaire. C'est pour cela que vous avez un double combat à mener au niveau européen. D'une part, vous devez préserver le budget de la PAC, qui est primordial et vital pour soutenir nos agriculteurs, et je sais que vous y travaillez. quand une norme nouvelle est appliquée en France ou, pire, quand un produit phytosanitaire est interdit ou va être interdit en France, il faut vous battre pour convaincre vos partenaires européens de suivre ces évolutions sociétales et de l'interdire aussi au niveau européen. Car c'est de cette façon que les agriculteurs français comprendront notre combat à tous pour une agriculture durable, une agriculture plus juste. Alors ensemble, dessinons l'agriculture durable que nous voulons. Car exiger toujours plus de nos producteurs et de nos filières sans soumettre nos voisins à la réciprocité conduisant aux mêmes pratiques vertueuses, c'est condamner demain l'ensemble des filières et notre indépendance alimentaire. Et après ? Nous importerons, comme nous le faisons déjà, des viandes sans savoir comment l'animal a été élevé et abattu, des fruits et légumes sans connaissance des modes de production, des produits alimentaires transformés dont nous aurons toutes les difficultés à connaître la traçabilité. Si nous voulons donner aux consommateurs la possibilité d'assumer leur responsabilité dans l'acte d'achat, il faut une traçabilité parfaite et un étiquetage précis. Pour que ce débat soit constructif, ne sortons pas des enjeux de ce texte les enjeux de santé, les enjeux environnementaux et, enfin, les enjeux économiques. À aucun moment nous ne pouvons traiter un enjeu sans les deux autres, car tous sont liés. Pour conclure, je dirai simplement que nous devons faire confiance à nos agriculteurs, qui ont bien compris les nouveaux défis.

entendre et à s'enrichir de l'expression de l'ensemble des acteurs concernés, de près ou de loin, par les activités agricoles et par les activités territoriales qui touchent à l'agriculture.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, annoncé comme issu des États généraux de l'alimentation, ce texte aurait dû afficher des ambitions pour le modèle agroéconomique de nos exploitations : revenus suffisants aux agriculteurs, alimentation saine et, bien sûr, respectueuse de l'environnement, compétitivité. Devant les très nombreuses rencontres et les centaines de contributions débattues par tous et partagées par le plus grand nombre, les agriculteurs, notamment, s'attendaient à un texte fondateur, novateur, consensuel et donnant confiance à l'avenir de cette filière économique de premier plan.

Trois préalables auraient dû transparaître dans la loi : harmoniser, notamment au sein de l'Union européenne, en évitant toute surtransposition des normes communautaires- c'était, faut-il le rappeler, un engagement du Président de la République République ; avant toute interdiction, s'assurer de disposer de solutions au moins aussi efficaces que les précédentes ; valoriser et soutenir les pratiques des agriculteurs qui ont accompli de multiples améliorations depuis des décennies, et ce bien souvent de manière volontaire. des agriculteurs font évoluer leurs métiers afin de protéger l'environnement, les milieux naturels et la santé des consommateurs. Elles ont été rendues possibles grâce à leur implication personnelle et à l'intégration de ces nouvelles pratiques dans leur plan de gestion et leur modèle économique. Je ne veux pas entrer dans le détail de ce texte- des collègues l'ont fait avant moi, et d'autres le feront encore -, mais plutôt exposer les solutions volontaires avancées par la filière agricole. Collectivement interpellés par les consommateurs sur leurs modes de production, ils continuent de répondre aux évolutions sociétales et portent l'ambition d'un « contrat de solutions ». Ce contrat, associant plus d'une Ce contrat, associant plus d'une trentaine d'organisations agricoles et de recherche, intègre toutes les productions, tous les territoires et toutes les filières. Il vise à développer l'innovation, le conseil, la formation et l'adoption d'alternatives de protection des cultures, afin de répondre concrètement aux attentes sociétales sur l'utilisation des produits phytosanitaires, tout en garantissant la compétitivité de la Ferme France. Avec ce « contrat de solutions », ils souhaitent être pleinement acteurs de la construction de modèles en sortant des interdits et en portant les performances économique, sociale, environnementale et sanitaire. Dans ce contrat important, plus de 250 solutions d'avenir ont d'ores et déjà été identifiées parmi les pratiques agronomiques, le numérique, l'innovation variétale, ou encore les techniques de pulvérisation et de mécanisation. Après ce projet de loi, il me semble important que l'État puisse s'engager avec la profession sur ce contrat qui doit être gagnant pour toutes les parties. Les agriculteurs sont prêts à vous le présenter, ils sont prêts à le mettre en oeuvre ; l'État est-il prêt à accompagner cette démarche ambitieuse ? L'État est-il déterminé à s'engager aussi, de manière pluriannuelle, sur les solutions efficaces et concrètes proposées par ces professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire ?

J'ai peur que la déception ne soit aussi forte que les espoirs suscités. Grâce au « contrat de solutions », l'occasion est donnée de remplir toutes les cases des objectifs environnementaux, sanitaires et économiques, et ce- c'est important -de manière volontaire

Les pesticides chimiques, qui ont imprégné notre environnement et notre agriculture, ont un impact sur la santé humaine. On observe une recrudescence des maladies environnementales et un effondrement de la biodiversité, en particulier des colonies d'abeilles. Mes positions sur ce texte, qui ne se veulent ni idéologiques ni dogmatiques, s'appuient sur ces deux axes : le « non-pesticides » et la promotion des agricultures vertueuses- je pense à l'agroécologie, dont l'agriculture biologique est le fleuron. J'ai été très déçu par l'examen du texte en commission des affaires économiques, mais j'espère encore que les débats en séance permettront au moins de revenir au niveau d'exigence de l'Assemblée nationale. Le retour en commission du 20 % de bio, ce matin,

Cette loi ne suffira pas pour retrouver des perspectives pour l'agriculture et l'alimentation. Il faudra une véritable planification sur le moyen et le long terme. Monsieur le ministre, si j'étais ministre de l'agriculture je proposerais : de mettre en place un plan réellement efficient de sortie des pesticides en soutenant fortement la conversion en bio bio ; d'encourager le retour à la polyculture élevage sur les territoires, avec des systèmes fourragers performants ; de réintroduire des ceintures maraîchères autour des centres urbains

enfin, pour assurer le renouvellement des générations et la formation des nouveaux agriculteurs. C'est véritablement un nouveau contrat de société que l'on doit mettre en place. Mais je ne suis pas ministre ... Ouf ! C'est pour cela que je me

des printemps de plus en plus silencieux. Notre responsabilité est de contribuer à offrir aux générations nouvelles des printemps joyeux et réenchantés ! La parole

Elle a permis de nourrir toute la population non seulement en quantité nécessaire, mais aussi en qualité sanitaire et nutritive. Ce qui en fait, n'ayons pas peur de le dire haut et fort, l'alimentation la plus saine et sûre au monde. C'est depuis quelques années, avec des médias à l'affût de tout événement croustillant susceptible de faire progresser leur audimat, et des personnes en recherche de notoriété, comme ce pseudo-agriculteur du Larzac, qui d'ailleurs ne l'a pas été longtemps, un courant de vents mauvais souffle sur l'image de notre agriculture. Cette même agriculture, plébiscitée hier par tous ces Français issus de familles agricoles sur deux ou trois générations, est aujourd'hui la cible de toutes les attaques. attaques. Attaques de tous ceux, passéistes et nostalgiques de l'agriculture de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, qui souhaiteraient, les dimanches ou pendant les vacances, avec tout le confort,

et favorisent l'importation de tonnes de denrées alimentaires produites dans des pays avec des règles environnementales et sanitaires aux antipodes des nôtres. Attaques par des politiques, plus du tout formés à la chose agricole et adeptes du renoncement perpétuel, qui ont pour seule devise, au lieu d'avoir le courage de regarder les choses en face, de céder lamentablement à la vindicte populiste de tous ces, anti-viande, altermondialistes. Alors, avec l'arrivée d'un Président-tout neuf, les agriculteurs, tellement accablés par tout cela et blessés dans leur chair, avec ce terrible sentiment d'injustice né du fait que, travaillant avec passion, ils ne récoltent que des critiques,

Nos agriculteurs y ont tellement cru qu'ils ont participé avec conviction aux États généraux de l'alimentation. Car, ne nous y trompons pas, ce qui caractérise les agriculteurs, c'est qu'ils croient que demain sera mieux qu'hier.

ces mêmes États généraux dans lesquels ils ont mis tant d'espoir, non seulement celui d'une juste valorisation financière de leur travail- qui peut nier la triste réalité du manque de revenu de la majorité de nos agriculteurs aussi, et peut-être surtout, l'espoir d'une reconnaissance nationale de leurs efforts, tant au cours des heures passées avec leurs animaux ou dans leurs champs que dans la technicité et la passion de produire au mieux une alimentation de qualité. Alors que nous discutons aujourd'hui au Sénat du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, que reste-t-il de cet espoir ? Rien ! Un véritable gâchis, dont vous êtes responsable, responsable de ne pas avoir pu tenir vos troupes à l'Assemblée nationale avec 2 700 amendements et 72 heures de défouloir durant lesquelles tout y est passé : caricatures, déformations, clichés. Tout cela téléguidé par un obscurantisme digne du Moyen Âge Le titre II du texte adopté par l'Assemblée nationale en est un exemple criant. Ce ne sera que des contraintes et des charges supplémentaires pour les agriculteurs

gagner la partie ? C'est d'une grande loi que l'agriculture avait besoin, une loi permettant de redonner de la fierté au paysan que je suis, et à tous les autres paysans de France,

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, vous qui avez fait un travail énorme avec les présidents de commission,

projet de loi. Monsieur le ministre, je crois que l'on peut partager vos intentions, que vous avez clairement exprimées. Nous sommes conscients que l'agriculture a besoin d'un électrochoc, qu'elle a besoin d'être accompagnée.

l'agriculture est dans une situation de concurrence mondiale. Aujourd'hui, les éleveurs bretons préfèrent acheter du blé d'Ukraine ... C'est vrai ! ... ou du soja d'Amérique du Sud pour engraisser leurs porcs.

La contractualisation entre agriculteurs, transformateurs et commerçants, par laquelle « le contrat et le prix associé seront proposés par celui qui vend

le biologique mondial ne vaut pas toujours le conventionnel français. Soyons prudents ! Si nous mettons

je vais concentrer mon propos sur un seul sujet, important, qui a fait l'objet d'âpres discussions lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytopharmaceutiques, au premier rang desquelles les agriculteurs. Le 1 février 2018, le Sénat a voté une proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation financé par les firmes elles-mêmes. Ce fonds permettra d'accompagner les victimes atteintes de maladies liées à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, en facilitant leurs démarches, en leur offrant un cadre global pour une plus grande égalité et en les indemnisant en réparation du préjudice intégral subi. Une mission interministérielle menée

que la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'usage de produits phytopharmaceutiques enregistrées depuis dix ans- moins de 1 000 cas -n'est pas à la hauteur de la réalité du nombre estimé de victimes potentielles. eux, cela peut s'expliquer par la difficulté à établir un lien de causalité entre la maladie et l'exposition à des substances nocives. Une estimation du nombre de victimes potentielles pour lesquelles il existe une présomption forte de causalité entre la maladie et l'exposition a été réalisée personnes seraient concernées sur dix ans, dont les deux tiers pour la maladie de Parkinson et un tiers pour les leucémies et les lymphomes. Monsieur le ministre, vous avez proposé à plusieurs reprises d'adapter le régime AT-MP pour mieux prendre en charge les victimes présumées des maladies liées aux produits phytopharmaceutiques, ce qui justifie, selon vous, de rejeter la création d'un fonds d'indemnisation. Pourtant, le rapport de l'IGAS, dont la rédaction est issue de trois ministères, y compris le vôtre, affirme en toutes lettres que des adaptations du régime AT-MP ne suffiraient pas pour indemniser l'ensemble des victimes présumées et qu'un fonds spécifique d'indemnisation s'avère pertinent. Alors, pourquoi s'obstiner à nier la vérité et ne pas permettre aux victimes d'obtenir une juste réparation ? Après le rapport de la mission d'information du Sénat de 2012, dont j'étais la rapporteur et Sophie Primas la présidente, qui a été voté à l'unanimité et dont des recommandations se sont déjà traduites dans la loi,

de réparer la souffrance de ces victimes que notre société n'a pas su, à ce jour, prendre en considération. Les victimes nous le demandent, elles attendent de nous que nous inscrivions maintenant, dans le

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, déception, déception, à laquelle s'ajoute l'amertume pour le monde agricole. Artifice, faiblesse du Gouvernement ? Peut-être. Trop grande détresse exprimée par toute une profession ? Sûrement. Qu'on en juge, mais le compte n'y est pas Être à la hauteur des attentes et des propositions des États généraux de l'alimentation n'est certes pas une tâche facile. Définir une nouvelle France agricole, tel est l'enjeu de ce projet de loi, qui s'appuie sur une déclaration solennelle du Président de la République. Hélas, nous en sommes très loin Je ne rappellerai pas l'état des lieux, fort bien exposé par les excellents rapporteurs du texte au nom de la commission des affaires économiques, Michel Raison et Anne-Catherine Loisier, dont le travail honore le Sénat. Un tiers de nos agriculteurs gagne moins de 350 euros par mois, 40 % des céréaliers affichent un revenu disponible négatif et le prix du lait stagne autour de 330 euros par tonne.

Il pense tout régler uniquement par le biais de modifications des contrats commerciaux entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Pour ma part, je souligne qu'il est indispensable qu'un tarif de base soit garanti aux producteurs de cultures végétales comme aux éleveurs, afin que le prix de vente de leur production ne soit jamais inférieur à leur prix de revient. Par ailleurs, la formation des prix, aussi nécessaire soit-elle, ne peut en aucun cas former le revenu des producteurs. Nous savons tous ici que, sans régulation des marchés au plan européen, l'ambition est vaine. Alors, attention aux désillusions ! Ne perdons pas de vue que le relèvement du seuil de revente à perte ou encore l'inversion de la construction du prix ne constituent pas des réponses à ces questions. La baisse des charges sociales, de plus en plus écrasantes, nous permettrait de sortir de ce marasme économique. Baisser l'ensemble des charges, monsieur le ministre, c'est permettre de réduire les coûts et de donner du à notre économie. Dans ce contexte, comment se dessine l'avenir, monsieur le ministre ? Je vous remercie de bien vouloir nous le préciser. L'une des pistes de transformation profonde de l'agriculture a été évoquée par le Président de la République : « Il faut doter la France d'un véritable projet agroécologique ». Est-ce suffisant ? Assurément non, si on ne tient tout simplement Les usages non alimentaires, dont les biocarburants, ont toute leur place dans ce dispositif. Ils peuvent contribuer à faire vivre de nombreux agriculteurs qui ont choisi de diversifier leur activité principale pour essayer de vivre décemment et échapper à un revenu qui peut faire d'eux des indigents. En outre, ce sont des ressources qui restent en France et peuvent prospérer. Les

la réduction des gaz à effet de serre, la baisse du CO2 et, à court terme, un mieux-être des populations en termes de santé publique, sans oublier notre indépendance énergétique, qu'il ne faut pas négliger. Or que fait actuellement le Gouvernement ? Plutôt que de favoriser la valorisation des coproduits de transformation agricole, acteurs majeurs des débouchés s'offrant à nos agriculteurs, il fait preuve d'un attentisme intenable et incompris.

Dois-je rappeler le sinistre exemple de l'usine de la Mède, qui n'est pas digne, monsieur le ministre, ou souligner que les mesures concernant l'anti-dumping sur l'huile de palme, qui ont été votées en décembre par le Parlement, ne sont toujours pas entrées en vigueur sept mois après ? Ce n'est pas normal ! Est-ce ainsi que le Gouvernement encourage nos agriculteurs qui font l'effort de se diversifier pour pouvoir enfin espérer vivre de leur travail et créer de la richesse pour la France ? Les efforts considérables déployés de leur part sont indéniables. Il faut les reconnaître et les encourager. À ce titre, je remercie la commission

Le Gouvernement a-t-il l'intention d'honorer ses promesses dans ce texte ? Le groupe Les Républicains, en ce domaine, ne peut pas se contenter d'un marché de dupes, car il souhaite profondément être au rendez-vous d'une nouvelle donne pour notre agriculture. Merci, cher collègue !

d'une prise en compte de la spécificité de l'agriculture dans les accords de libre-échange, notamment par l'insertion de la notion de réciprocité. Ce travail va dans le bon sens, mais pour protéger efficacement notre agriculture et notre souveraineté alimentaire, nous devons aller C'est pour cela que nous proposons d'instaurer une véritable exception agricole lors des négociations d'accords de libre-échange sur le modèle de l'exception culturelle. Cette proposition avait déjà été défendue par plusieurs personnalités, dont notre actuel ministre de la transition écologique et solidaire dans une tribune en 2016. La nourriture est un besoin humain et, à ce titre, elle ne peut pas être considérée comme une marchandise comme les autres. Notre souveraineté alimentaire ne peut en aucun cas constituer une monnaie d'échange. Le XXIsiècle présente des défis climatiques et alimentaires, que nous avons le devoir et la responsabilité de relever pour préserver notre planète et ses ressources. Or les nouveaux traités bilatéraux, à l'exemple du CETA avec le Canada et de bien d'autres, présentent des risques importants en termes économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux et favorisent l'abaissement des normes sur ces sujets. Par exemple,

Dans la perspective des engagements de la France à lutter contre le changement climatique et au nom de la défense de notre souveraineté alimentaire, cette proposition entend reconnaître une exception agriculturelle dans les échanges internationaux. Cette démarche permettrait de déverrouiller les négociations des autres volets commerciaux des traités multilatéraux, aujourd'hui enrayées par des accords bilatéraux.

le fait que l'agriculture ne saurait être appréhendée comme un secteur économique ou une marchandise. Les États généraux de l'alimentation nous ont rappelé une chose essentielle : notre modèle agricole est unique, notre agriculture est performante et nous souhaitons tous en préserver les spécificités qui en font la richesse. Pour l'instant, est celui de la mondialisation, de la libéralisation des échanges et de la concurrence économique. Dans ce contexte, nous devons mettre en place des garde-fous dans un certain nombre de secteurs stratégiques. L'agriculture fait partie de ces secteurs, car elle nous renvoie à la question fondamentale de notre souveraineté alimentaire, sujet particulièrement important à l'heure des changements climatiques et des inquiétudes qui en découlent. C'est en outre un marqueur culturel fort, que chaque pays devrait avoir à coeur de défendre. Dans les années quatre-vingt, la France obtenait la reconnaissance d'une « exception culturelle ». Nous pensons que, trente-cinq ans plus tard, il est temps de faire de même pour notre agriculture. Comme le rappelaient les auteurs d'une tribune parue en 2016 en faveur de cette démarche, et dont M. Hulot était signataire, la reconnaissance d'une « exception agriculturelle » dans les traités commerciaux permettra de progresser sur les autres volets commerciaux des négociations multilatérales et renforcera la gouvernance mondiale qui en résulte. Mes chers collègues, ce projet de loi se fixe pour objectif d'augmenter le revenu des agriculteurs, et nous aurons l'occasion de discuter de sa réelle capacité à le faire, mais, tant que la question de la préservation de notre modèle et de nos agriculteurs face à la concurrence internationale ne sera pas traitée-

à dire que les missions de la politique agricole, telles qu'elles résultent de l'article 11 , incluent déjà la promotion de l'indépendance alimentaire de la France, la préservation de son modèle agricole et l'exigence de réciprocité dans tout accord de libre-échange.

du Gouvernement ? Le Gouvernement, vous le savez, est totalement mobilisé pour garantir l'égalité de concurrence entre les producteurs français et leurs homologues européens. Nous travaillons beaucoup dans ce sens. Cependant, une « exception agriculturelle » française qui serait conçue sur le modèle de l'exception culturelle, c'est-à-dire qui soustrairait le secteur agricole français du cadre commercial multilatéral, n'est pas envisageable. En effet, une telle attitude exposerait la France à des sanctions internationales, d'abord dans le cadre de l'OMC, et priverait priverait nos exploitants agricoles de débouchés économiques importants. En outre, la France perdrait le bénéfice du cadre de régulation des échanges agricoles et de protection des standards internationaux, notamment sanitaires, auxquels nous sommes

de la façon dont ils vont se dérouler. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions commencé le débat sur la loi Asile et immigration par les quotas ... Aujourd'hui, ces amendements nous donnent l'occasion

l'environnement, la biodiversité, l'aménagement de l'espace, l'aménagement du territoire. Elle a aussi un rôle culturel, éducatif ; elle joue sur le plaisir et a même parfois un rôle philosophique, comme l'affirmait Brillat-Savarin : « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai

l'exception agriculturelle. Voilà 15 000 ans, c'est grâce à l'instauration de l'agriculture que notre civilisation a pris un nouveau cours. Je ne suis pas loin de considérer qu'aujourd'hui nous devons nous reposer la question de la centralité de l'agriculture dans nos sociétés, dans notre civilisation.

Tel n'est pas été le cas dans tous les autres pays d'Europe et du monde. Il n'y a pas besoin de se poser des questions sur le libre-échange ; commençons par avoir une vision claire et précise de ce que l'on veut faire de notre agriculture. Soutenons-la quand elle a besoin d'être soutenue,